La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 16 décembre 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Stéphane Bonduel, qui fut sénateur de la Charente-Maritime de 1980 à 1989, et Louis-Ferdinand de Rocca Serra, qui fut sénateur de Corse-du-Sud de 1994 à 2001. Mes chers collègues, au vu de l'évolution de la situation sanitaire et après concertation du président du Sénat avec les questeurs, les présidents de groupe et les présidents de commission et de délégation, il a été décidé de ne pas rétablir de système de jauge pour la séance publique et pour les réunions de commission et de délégation. En revanche, les commissions et les délégations ont de nouveau la possibilité d'organiser leurs réunions plénières selon un schéma mixte le présentiel en principe, mais la faculté de participer à distance, sans toutefois la possibilité de voter pour ceux de nos collègues utilisant la visioconférence. Sur la proposition de M. le président du Sénat, nous pourrions également suspendre l'application de l'article 23 de notre règlement, relatif aux présences en séance publique et en commission, jusqu'à la suspension de nos travaux, à la fin Aucune retenue ne serait donc effectuée en application de cet article au terme de la période de référence de quatre mois initialement retenue. Il n'y a pas d'opposition ? Il en est ainsi décidé. Je vous rappelle enfin que le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs s'exprimant à la tribune. J'invite par ailleurs chacune et chacun à veiller au respect des gestes barrières,

de l'ordre du jour du jeudi 6 janvier la séance de questions orales et a sollicité du Sénat l'inscription, le jeudi 6 janvier, l'après-midi et le soir, du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, le vendredi 7 janvier, l'après-midi et le soir, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de l'éventuelle commission mixte paritaire sur ce texte. Le texte n'ayant pas été transmis cette nuit par l'Assemblée nationale, son inscription à l'ordre du jour sera soumise ultérieurement au Sénat. Par ailleurs, en raison de la demande du Gouvernement, il était envisagé de soumettre au Sénat les modifications suivantes : d'une part, l'avancement à la reprise de ce soir du débat sur la politique mise en place par le Gouvernement pour conforter la souveraineté maritime française sur les océans, initialement prévu le jeudi 6 janvier après-midi, avec un délai d'inscription de parole aujourd'hui à d'autre part, l'avancement au jeudi 6 janvier, à dix heures trente, du débat sur le thème « Le partage du travail : un outil pour le plein emploi ? », ainsi que du débat sur la sûreté des installations nucléaires, initialement prévus l'après-midi. Après consultation des groupes politiques, nous pourrions procéder à ces modifications de notre ordre du jour. Il n'y a pas d'opposition ? ... Il en est ainsi décidé. Enfin, le Gouvernement a demandé dans sa lettre d'ordre du jour l'inscription d'une séance de questions orales le mardi 25 janvier au matin, en remplacement de celle de ce jeudi. Acte est donné de cette demande. demande. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires économiques a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

Je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé d'expérimenter une proposition du groupe de travail sur la modernisation des méthodes de travail du Sénat. En application de cette proposition, le groupe Les Républicains disposera d'un temps de présentation de huit minutes, le Gouvernement lui répondant pour une durée équivalente. Lors du débat interactif, le Gouvernement aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de répondre à une réplique pendant une minute ; l'auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a cinq ans, le candidat Emmanuel Macron promettait un choc d'offre afin de faire baisser les prix du logement. Il promettait également de construire 60 000 logements étudiants et de répondre aux besoins des ménages aux revenus les plus modestes. Aujourd'hui, à l'approche d'échéances essentielles pour notre pays, il est temps de faire le bilan du quinquennat en matière de logement et de politique de la ville. Force est de constater que le choc d'offre a laissé place à l'aggravation de la crise du logement, l'espoir pour les plus modestes à un horizon bouché et l'effacement des ghettos à la persistance des barrières à l'intégration. Face à ce bilan, que nous dénonçons, le groupe Les Républicains veut formuler de véritables propositions alternatives pour notre pays et pour tous les Français. En effet, cinq ans après ces promesses, comment ne pas être frappé par l'inquiétude des Français ? Les prix des logements s'envolent, au point de devenir inaccessibles pour nombre de nos concitoyens. Il en est de même des prix de l'énergie, qui pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat. Dès lors, malgré les discours officiels, les Français ont le sentiment de se précariser et même d'être déclassés. Le logement, symbole de sécurité pour chaque famille, est au coeur de leurs préoccupations. Sortir du logement social, devenir propriétaire, acheter une maison avec jardin comme l'ont fait leurs parents avant eux sont autant de projets qui deviennent des chimères.

Si le décalage est si grand entre les promesses et la réalité vécue par les Français, c'est bien à cause d'un quinquennat qui, en adoptant une vision technocratique, a délibérément fait du logement des plus modestes un poste d'économies budgétaires.

Action Logement a été menacé de démembrement et ponctionné de plus de 2 milliards d'euros. Malgré la prolongation de la loi relative de tardives ambitions en matière de logement social, la réalité des faits passés et la vision macroéconomique de l'exécutif ne peuvent que confirmer nos inquiétudes. ce que nous constatons, c'est la volonté persistante de remettre en cause le modèle français du logement social et de prolonger la rupture qui s'est produite en 2018 : « la mutation majeure du logement social solide vers le logement abordable liquide », c'est-à-dire un logement social réservé aux populations les plus fragiles et financé, soit par les ventes de logements, soit par le marché, tandis que ses ressources propres- livret A et 1 % logement -seraient partiellement réduites ou réallouées. La dépense nationale pour le logement, supposée inflationniste, continuerait quant à elle de baisser.

Au mieux, 30 000 logements étudiants seront construits sur les 60 000 promis. Certes, la crise sanitaire a eu un impact, de même que les élections municipales, mais ces éléments conjoncturels ne dédouanent en aucun cas le Gouvernement de sa responsabilité.

Le rapport Borloo proposait une vision de société ; il a été rejeté. Par deux fois, les maires des quartiers prioritaires ont dû lancer un appel au secours au Président de la République pour ne pas être oubliés.

Face à ces résultats qui désespèrent les Français, je tiens à le réaffirmer : une autre politique était et est toujours possible. Le plan de relance a été une occasion manquée de relancer la construction. concerne le logement social, il était possible de redonner de l'oxygène aux bailleurs, par exemple en rétablissant le taux de TVA à 5,5 % pour toutes leurs constructions, à tout le moins

C'était aussi le bon moment pour s'attaquer au statut du bailleur privé. À force de considérer l'investisseur immobilier comme un rentier improductif et non comme un entrepreneur en logement, on a obéré durablement le logement locatif.

La multiplication des normes pèse sur le coût de la construction. C'est en écoutant les acteurs de terrain que nous parviendrons à cette simplification. Ensuite, et surtout, il faut rétablir la fluidité du parcours résidentiel. Les Français ne souhaitent pas rester locataires toute leur vie, dans le parc privé ou dans le parc social. L'accession à la propriété est une aspiration légitime, qui doit être soutenue. C'est un aspect central de l'ascenseur social. Il faut lever les obstacles qui l'empêchent. Valérie Pécresse a récemment souligné l'injustice des primes d'assurance emprunteur pour les personnes séropositives ou celles qui ont été atteintes d'un cancer.

pour mettre fin à la concentration de la pauvreté et ouvrir les villes concernées à une plus grande diversité. Nous le savons bien : c'est cette concentration qui fait le lit de toutes les difficultés. Il nous faut aussi revenir à un modèle du logement social ouvert aux classes moyennes Ces Français ont le droit d'habiter près de leur lieu de travail. Demain, ils seront autant d'exemples pour l'intégration. Il nous faut enfin, comme l'a proposé l'institut Montaigne, créer une ANRU des habitants à côté de celle des bâtiments, pour accompagner les populations de ces quartiers, souvent animées d'un véritable esprit d'entreprise, vers la réussite économique et l'intégration dans la République. Mes chers collègues, l'inaccessibilité du logement est un facteur majeur de précarisation et de blocage de l'ascenseur social. Chaque Français a pour aspiration d'offrir un toit à sa famille. Ayons l'ambition de proposer et de mettre en oeuvre les réformes nécessaires pour répondre à ce besoin essentiel, pour en faire un

alors que la demande est toujours forte dans les grandes villes, la construction de nouveaux logements ne suit pas. Or ne pas répondre à ce besoin, c'est organiser l'éviction des plus pauvres en périphérie, travail une partie de la population active et accroître le recours aux transports individuels. Cette situation a encore été accentuée par la crise sanitaire que nous traversons.

à saluer les sénateurs Estrosi Sassone, Marchand, Lienemann et Martin, qui ont représenté la Haute Assemblée au sein de cette commission. Les recommandations émises sont très claires : État, collectivités, promoteurs, bailleurs sociaux, mais aussi citoyens, nous devons tous réhabiliter l'acte de construire. Le Gouvernement a repris plusieurs propositions de cette commission, comme la signature, dans les territoires tendus, de contrats de relance du logement : au total, 175 millions d'euros du plan France Relance sont mobilisés à cette fin. Ils constituent le volet « logement » des

Ces efforts pour la construction et la mobilisation du parc existant se doublent d'un soutien à la production équilibrée de logements sociaux dans les territoires. Ainsi, ce gouvernement a engagé la pérennisation de la loi SRU avec le projet de loi 3DS, adopté en première lecture au Sénat. Nous saluons le travail accompli en ce sens par Dominique Estrosi Sassone et Valérie Très bien ! Cet exemple le confirme une nouvelle fois : le Gouvernement est pleinement mobilisé en faveur du logement abordable. En cohérence, nous agissons de manière déterminée dans les territoires fragilisés de la politique de ville. soyez assurés que n'avons pas perdu une once de notre ambition pour la réussite des habitants de ces territoires. Il me paraît bon de le rappeler : dès 2017, le Président de la République a décidé, non seulement de doubler l'enveloppe de l'ANRU,

d'euros engagés. Ce sont là autant d'actions menées et renforcées, à la suite de la crise sanitaire, pour remettre les territoires au coeur de notre pacte républicain. À l'issue du comité interministériel des villes du 29 janvier 2021, nous avons tenu à aller plus loin

permis de débloquer des dossiers ankylosés depuis de trop nombreuses années. Nous agissons aussi pour la tranquillité des habitants. C'est l'une des principales préoccupations de nos concitoyens et c'est aussi la nôtre. Nous agissons pour réaffirmer l'autorité en créant 1 200 postes de policiers et de gendarmes dans 62 quartiers de reconquête républicaine et en augmentant les moyens accordés à la justice, notamment en renforçant la justice de proximité pour traiter la délinquance, la criminalité et les différentes formes de séparatisme qui rongent le quotidien des habitants. En même temps, nous travaillons à la prévention du passage à l'acte en créant 45 bataillons de la prévention. regroupent 600 éducateurs et médiateurs formés pour aller vers les jeunes et remobiliser ceux qui sont les plus éloignés de ce qui fonde notre pacte républicain, à savoir la citoyenneté, l'emploi et l'école. Nous voulons assécher ce qui peut constituer un vivier de recrutement

est un levier incontournable pour l'attractivité des territoires, les emplois et la qualité de vie. Je pourrais vous parler encore longtemps des autres actions que nous mettons en place, comme les maisons France Services, le dispositif Nature en ville ou les quartiers productifs, mais le temps m'est compté. Cela étant, je ne doute pas que nous reviendrons au cours du débat sur ces initiatives fondamentales. Notre ambition reste

votre collègue chargée du logement a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques mois en affirmant : « Le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène dans une impasse. » L'habitat individuel étant plébiscité par plus de 80 % des Français, cette phrase a pu choquer certains. Toutefois, la crise écologique et la crise que connaît notre pays en matière de logement nous poussent à nous interroger sur les modèles qui régissent notre conception de l'habitat. Sur les 37 millions de logements existants, 55 % sont des logements individuels. Or nos collectivités territoriales se trouvent confrontées à un double impératif concilier le besoin croissant de logements et la préservation de l'environnement, notamment en respectant l'objectif de « zéro artificialisation nette » des sols. Dans certains territoires, cette équation se solde par des prix de l'immobilier qui flambent et qui représentent une charge intolérable pour les ménages. Les 10 % des foyers les plus modestes consacrent près de la moitié de leur budget au logement. Dans les villes, les entreprises peinent à recruter les travailleurs clés qui font tourner l'économie, mais ne peuvent plus habiter sur place. Aussi, certaines collectivités font le choix de construire la ville sur la ville, c'est-à-dire de construire sans s'étaler.

la maison individuelle représente encore 40 % des logements autorisés, et une large majorité des permis de construire se situent dans les couronnes des pôles urbains. Dans le même temps, les centres-bourgs des petites villes se vident de leurs habitants et, dans les campagnes, on constate un quasi-gel des permis de construire. Ma question est la suivante : quelles sont les intentions du Gouvernement pour répondre à la crise du logement, c'est-à-dire construire plus, mais surtout construire mieux, tout en restant à l'écoute des attentes des Français quant à leur parcours résidentiel ?

nous pouvons aussi répondre à la demande en utilisant le parc déjà construit : c'est tout le sens de notre politique de rénovation énergétique des bâtiments. D'ailleurs,

Or cette ambition n'a jamais vu le jour, d'abord en raison d'un désengagement manifeste de l'État envers une politique pourtant essentielle pour la cohésion nationale. Il suffit de rappeler que l'initiative Coeur de quartier, annoncée au mois de juillet 2018 2018 n'a jamais vu le jour alors qu'elle était censée répondre au rapport Borloo. Mieux : interrogé par des maires à ce sujet cet automne, le Premier ministre n'en avait jamais entendu parler Seules des mesures éparses ont pu être engagées, très souvent sur l'initiative des villes et sans accompagnement de l'État. Le système des appels à projets pèche par son manque d'efficacité. La méconnaissance des procédures et les retards dans la constitution des dossiers entraînent une précarité des financements et des inégalités entre les communes. C'est souvent « premier arrivé, premier servi Madame la ministre, nous ne pouvons que constater l'absence totale d'une vision gouvernementale de la politique de la ville. La sanctuarisation des crédits fait chaque année l'objet d'angoisses de la part des élus et des acteurs de la rénovation urbaine, comme d'âpres négociations au Parlement. Certes, les crédits du plan de relance sont arrivés dans ces territoires, mais de façon très inégale et toujours précaire. Quel avenir pour des dispositifs efficaces comme Quartiers d'été et Vacances apprenantes ? Quel avenir pour les postes créés, par exemple pour la mise en place des bataillons de la prévention ? Madame la ministre, malgré le plan de relance et le budget 2022, les maires dénoncent une non-assistance à territoires en danger et un décrochage de la République. Qu'avez-vous à répondre à cela ?

Oui, madame la sénatrice, le visage de nos quartiers change, et il change avec les élus locaux ! Ce à quoi nous travaillons avec eux, ce sont non seulement des dispositifs, mais aussi une nouvelle manière de faire, une nouvelle forme de contractualisation qui permet à l'action de l'État de gagner en agilité et en efficacité,

ouvert une concertation à grande échelle impliquant les associations d'élus et les associations présentes sur le terrain, pour pérenniser ces dispositifs et réfléchir à la meilleure façon d'intervenir dans nos quartiers, particulièrement dans les territoires les plus fragiles.

Votre bilan n'est pas bon, madame la ministre. Vous n'avez aucune ambition pour la politique de la ville. Les dernières réponses non pérennes apportées en la matière n'y changeront rien.

en périphérie immédiate de la ville de Lille, commune qui compte deux quartiers inscrits en géographie prioritaire de la politique de la ville. Comme nombre de mes collègues, j'ai été régulièrement confronté à une équation impossible à résoudre- elle n'est d'ailleurs toujours pas résolue -, celle du nombre de demandes de logements face au taux de vacance dans le patrimoine locatif, notamment dans celui des bailleurs sociaux. La construction de logements est bien évidemment une réponse à ce problème. La commission pour la relance durable de la construction de logements, sous la présidence de M. François Rebsamen, a remis les deux tomes de son rapport, lequel formule nombre de propositions visant à simplifier l'acte de construire et à accélérer les procédures d'urbanisme. Il me semble cependant qu'une partie de la réponse aurait pu et pourrait encore être apportée si un véritable travail d'inventaire était effectué et si des moyens étaient mis en place pour régler, ou tenter de régler, le sujet de la concordance entre typologie du logement et composition de la cellule familiale. familiale. Pour préparer ce débat, je me suis rapproché d'un bailleur social nordiste, aujourd'hui propriétaire de près de 73 000 logements et qui loge 171 000 personnes- soit un ratio de 2,1 personnes par logement, ce qui est fort peu au regard de la typologie des logements proposés. Combien d'exemples avons-nous dans nos communes et dans nos QPV de logements de type 4 ou 5, hier encore occupés par une famille de quatre ou cinq, voire six personnes, et qui, au fil des années, ont vu leurs occupants partir

inciter les occupants à changer de logement pour une typologie plus adaptée, mais chacun sait bien qu'il est plus que difficile de quitter son logement, voire son quartier, dans lequel toute une vie a pu s'écrire. vous savez comme moi que les bailleurs sociaux ont bien des missions à remplir, notamment pour faire du vivre ensemble une réalité dans nos QPV, et que la question de l'adéquation du logement avec le nombre d'occupants ne peut être résolue faute de moyens et de dispositifs financiers, ces derniers restant à imaginer. Madame la ministre, ma question est simple : pouvez-vous me dire si cette piste est aujourd'hui à l'agenda ? La parole est à Mme la ministre

d'abord, elle a généralisé la gestion en flux des contingents de réservataires dans le parc social pour les bailleurs. Cette disposition vise à améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande et à élargir la palette de choix pour les ménages, en fonction de leurs besoins. Cette loi a

procède ensuite, avec le locataire, à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel. Toutefois, la situation de nos QPV mérite une attention particulière, vous l'avez souligné, monsieur le sénateur. Il est important de maintenir dans ces parcs sociaux des occupants historiques aux revenus plus élevés que ceux des nouveaux entrants, afin de favoriser le vivre ensemble. C'est pourquoi les dispositions législatives qui suppriment le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locataires en situation de sous-occupation dans les zones tendues ne s'appliquent pas dans les QPV. L'enjeu est plutôt de stabiliser l'occupation et de redonner de l'attractivité à ces quartiers et au patrimoine social, en le réhabilitant. Cela permettra aussi de répondre au nombre parfois important de refus dont font l'objet les propositions de logement dans certains QPV. Afin de faciliter la mobilité dans le parc social, nous continuons à encourager les bonnes pratiques et les démarches Je pense à des actions à l'initiative des organismes de logement social ou de réservataires, par exemple dans le cadre de démarches interbailleurs, à l'instar de la bourse Échanger Habiter en Île-de-France. Vous le voyez, monsieur le sénateur : le Gouvernement est pleinement

en économie, il est une loi intangible : la rareté crée la valeur. Quand il y a abondance, les prix baissent ; quand il y a carence, les prix augmentent. Le foncier n'échappe pas cette règle. Cependant, il se distingue par une spécificité notable : ce sont les pouvoirs publics qui décident de sa disponibilité sur le marché.

la stratégie que le Gouvernement a adoptée restreindra drastiquement les surfaces constructibles. Mécaniquement, il est facile d'anticiper une hausse spectaculaire des prix dans les prochaines années. Cette donnée est évidemment clé pour rebâtir une politique du logement ambitieuse. Comment faciliter l'accès au logement, que ce soit par l'offre de logements sociaux ou par l'accès à la propriété, dès lors qu'une pénurie s'annonce sur la première des matières, à savoir le foncier disponible ? Il faut ajouter à cela toutes les contraintes légales qui s'accumulent pour les constructeurs. Je pense évidemment aux obligations environnementales, notamment à la loi sur l'eau et les milieux aquatiques qui complique les initiatives de nos entrepreneurs. Il faut également ajouter à cela l'augmentation des coûts liée à la réglementation thermique 2020, à laquelle les entrepreneurs peinent encore à s'adapter. Dans le même temps, la main-d'oeuvre demeure très chère les prix des matériaux s'envolent. Madame la ministre, comment le Gouvernement compte-t-il enrayer cette mécanique implacable du renchérissement ? Comment garantir aux Français des logements abordables ? La parole est à Mme la ministre

de front ces deux objectifs, car il est essentiel de réduire le rythme auquel nous bétonnons nos sols tout en construisant mieux, là où se trouve le besoin de logements. Je rappelle que l'objectif « zéro artificialisation nette » doit être atteint en 2050, de façon progressive, et non pas dès à présent. La loi Climat et résilience, qui fixe la trajectoire de réduction du rythme d'artificialisation des sols, permet, en l'état, d'avoir 140 000 hectares constructibles pour les dix prochaines années sur le territoire national. est très important, vous en conviendrez. Vous mentionnez également les coûts supplémentaires qu'induirait la nouvelle réglementation environnementale 2020 et le temps d'adaptation nécessaire pour Je rappelle que cette réglementation a fait l'objet d'une concertation intense avec l'ensemble des professionnels. Les coûts induits sont très faibles : environ 3 % pour le jalon 2022. à mettre en regard des économies générées sur les factures d'énergie des ménages. Enfin, l'accès au logement abordable est une priorité du Gouvernement. Nous avons pris plusieurs mesures historiques afin d'accompagner le secteur du logement, à court terme face à la crise sanitaire, mais aussi à moyen terme,

Marta de Cidrac. Madame la ministre, la crise du logement est une crise tout aussi quantitative que qualitative. Il y a six mois, vous avez lancé « Mieux habiter demain en ville », dont l'un des axes de travail était consacré à la qualité du logement. À cette occasion, les résultats de l'enquête Qualitel ont été publiés. Cette enquête pointe une baisse des hauteurs sous plafond, le manque de rangements et le manque d'espaces extérieurs. Une table ronde sur la qualité du logement a donné lieu à la présentation d'un référentiel, qui met en avant un critère essentiel : une surface minimale par type de logement. Ce référentiel souligne également les questions de volume, d'accès à un espace extérieur et de qualité de ventilation- preuve que la qualité du logement est un sujet multifactoriel. Au-delà de la qualité du neuf, l'amélioration de l'existant reste un véritable problème. Plusieurs mesures ont été prises, mais il manque un mouvement global allant au-delà des efforts individuels. Récemment, plusieurs instances ont fait des propositions pour mutualiser les efforts de rénovation à l'échelle des copropriétés, voire des quartiers, afin de diminuer les coûts et de massifier les gains des rénovations- propositions que vous regardez, je l'espère, avec intérêt. Aussi, madame la ministre, quelles suites comptez-vous donner au référentiel du logement de qualité ? Comment faciliter les dynamiques collectives de rénovation de l'existant ? La parole est à Mme la ministre

Se sentir bien chez soi, alors que l'on est amené à y passer de plus en plus de temps, à y travailler, à y vivre différemment, doit être un enjeu majeur pour nos politiques publiques. C'est pour cela que la ministre Emmanuelle Wargon a confié à François Leclercq et Laurent Girometti la mission de construire un référentiel de la qualité d'usage du logement, conviction que nous devions nous intéresser à la vie dans les logements, mais qu'il fallait le faire de façon différente, sans imposer de nouvelles normes réglementaires. L'État a choisi d'accompagner concrètement cette démarche. Certains critères du référentiel seront ainsi utilisés pour le paramétrage du dispositif Pinel à compter de 2023, notamment la présence systématique d'un espace extérieur ou la double exposition à partir du T3. Les critères de qualité doivent également trouver une traduction opérationnelle dans nos projets. La qualité du logement, c'est aussi l'affaire des maires. Le ministère du logement est ainsi plutôt favorable aux chartes locales de qualité mises en oeuvre par certaines collectivités, à condition de construire plus, de construire mieux, et non de construire moins. Nous voyons beaucoup d'exemples vertueux dans certaines villes, comme la charte récemment signée par la ville de Nice. Il est nécessaire d'engager un travail de fond sur ces solutions locales, afin d'identifier les bonnes pratiques, mais aussi de pointer leurs écueils. Le référentiel sur la qualité d'usage du logement pose aussi les bases de ce travail. Vous le voyez, madame la sénatrice, le Gouvernement soutient l'amélioration de la qualité des logements, car il s'agit de l'un des leviers à actionner pour relancer la construction et rendre l'habitat collectif

Il n'aura pas fallu moins qu'un appel très solennel de nombreux maires pour qu'une petite partie du plan de relance soit fléchée vers ces quartiers. Il aura aussi fallu, d'ailleurs, dès le début du quinquennat, en 2017, un appel de maires

toute la politique qui est menée parallèlement. La politique du Gouvernement en faveur des quartiers ne se limite absolument pas au plan de relance ! Quand vous parlez de la réhabilitation des quartiers, vous occultez totalement

soyez sûre que nous sommes, nous, au rendez-vous dans ces quartiers prioritaires. Je me demande si la présidente de la région Île-de-France est autant au rendez-vous dans ces quartiers et ces territoires que, nous, nous ! Ne nous demandez pas de nous substituer à la compétence de la présidente de la région Île-de-France. L'État intervient aux côtés des élus. C'est ce que nous faisons dans le Val-de-Marne et sur le territoire national. Taillé-Polian. Je ne dirai certainement pas que Mme la présidente de la région Île-de-France tient ses promesses et fait ce qu'elle devrait faire pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser cet argument pour justifier votre absence de politique Aujourd'hui, et depuis bientôt cinq ans, des associations sont en grande souffrance du fait de la fin des contrats aidés. Votre politique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, comme dans toute la France, d'ailleurs, conduit à une intensification de la pauvreté. Or où sont logés la plupart des gens en situation difficile dans notre pays, sinon dans les QPV ?

en particulier la hausse démesurée des dépenses de logement. Les loyers ont augmenté plus que l'inflation et plus que le niveau de l'évolution des revenus.

M. Macron voulait s'attaquer à la rente. Pourquoi ne s'est-il pas attaqué à la rente foncière, qui prend de la valeur sans que les gens fournissent des efforts ? Le Gouvernement n'a rien fait pour réduire ces divergences dangereuses entre l'évolution des prix du logement et les revenus. Au contraire, il les a laissées s'accroître. Pis encore, il a baissé la part des APL

précieux aux collectivités souhaitant s'engager dans une politique de maîtrise foncière et de régulation des coûts. À cela s'ajoute enfin le développement du bail réel solidaire (BRS) porté par les offices fonciers solidaires (OFS), que nous renforçons encore dans le projet de loi 3DS. En distinguant la propriété foncière et la propriété bâtie, en encadrant les prix de cession des des logements, le BRS propose aussi une réponse innovante et adaptée. En près de cinq ans, 71 OFS ont été agréés et une trentaine devraient l'être à court terme. Plus de 500 logements ont été déjà commercialisés en BRS, et ce parc dépassera probablement les 10 000 unités en 2024. Vous le voyez, madame la sénatrice,

Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la ministre, alors que rien ne le laissait prévoir dans son programme, le Président de la République a appliqué des coupes budgétaires dans le secteur du logement, se concentrant particulièrement sur le logement social et sur l'accession sociale à la propriété.

qu'ont connues les acteurs de ce secteur : prélèvements sur les budgets d'investissement des organismes HLM, suppression de l'aide aux maires bâtisseurs ainsi que de l'aide à l'accession, restriction du prêt à taux zéro (PTZ), tensions économiques générées par la crise sanitaire et les élections municipales. à la méthode mise en oeuvre : les bailleurs sociaux n'ayant pas été consultés préalablement, ils n'ont pas pu s'adapter et anticiper. Ils ont donc subi ces restrictions budgétaires qui ont largement affecté leurs capacités d'investissement et de production.

et 2019. Où se situe donc la baisse de logements autorisés, selon vous ? Vous avez appelé l'attention du Gouvernement sur la situation du logement dans les outre-mer, particulièrement sur la question de l'accès au logement social à La Réunion. Permettez-moi de rappeler que le plan Logement outre-mer 2019-2022 y a été décliné après concertation avec plus de 250 participants. Ce plan a un objectif moyen annuel de production de 2 000 à 2 500 logements locatifs sociaux, du même type, ainsi que d'amélioration de 400 logements privés indignes ou insalubres, afin de répondre aux objectifs de croissance démographique d'ici à 2035. Vous abordez également la question de l'inflation réglementaire.

propres. À La Réunion, une réflexion a été engagée avec les acteurs de la filière de la construction sur la maîtrise des coûts sans renoncer à la qualité des logements. Il s'agit de trouver des solutions et des réponses locales, avec les acteurs de terrain. Au-delà de la question de la relance du logement social et de la maîtrise des coûts, passe non pas par une qualité moindre, mais par une incitation plus importante des élus à délivrer des permis de construire, les contrats de relance du logement ont été mis en place sur les crédits du plan France Relance. C'est la raison pour laquelle, s'agissant des agréments délivrés à compter de 2021 et jusqu'à la fin du mandat municipal

Ces dossiers me semblent démontrer notre capacité à développer des projets ambitieux dans le cadre de démarches partenariales associant l'État, les collectivités locales et les bailleurs sociaux. Pour autant, bien que décisifs, ces projets ne suffisent pas à masquer la défaillance des politiques de logement social et la réalité des chiffres. Dans le Gard, avant même la crise sanitaire, la production de logements sociaux a ainsi été divisée par deux entre 2018 et 2019. Madame la ministre, je ne reviendrai pas sur la baisse surprise des aides personnalisées au logement (APL) dès 2017, mais il est clair qu'en matière de logement votre gouvernement a fait de véritables choix politiques.

Alors que le Président de la République affirmait sa volonté de créer un choc de l'offre, on a vu se multiplier les dispositifs donnant des signaux totalement inverses : fragilisation des organismes HLM au travers de la relèvement du taux de TVA pour les logements sociaux, restriction du champ d'application des prêts à taux zéro, suppression de l'APL accession, etc. Selon la Fondation Abbé Pierre, Selon la Fondation Abbé Pierre, au cours des cinq dernières années, plus de 10 milliards d'euros d'économies ont été réalisés au détriment du logement des Français les plus modestes. Aussi ma question est-elle simple, madame la ministre : comment expliquer un tel décalage entre l'objectif affiché et les dispositions prises ? Comment revendiquer un choc de l'offre visant à tasser les prix et, « en même temps », ponctionner de la sorte la capacité d'investissement des bailleurs sociaux ?

des mesures de soutien massif ont été prises dans le cadre du pacte conclu en 2019 avec le secteur, comprenant notamment le gel, puis la révision de la formule de calcul du livret A et un soutien accru de la banque des territoires et d'Action Logement.

pour tous les logements sociaux agréés entre 2021 et 2026. Au total, les études perspectives de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) démontrent que la situation financière du secteur est très solide : elle est comparable à celle de 2014. Ce quinquennat n'aura donc pas du tout sonné le glas

Meurant. Madame la ministre, « décevante et coûteuse », voilà comment la Cour des comptes, qualifie la politique du logement en France. Pourtant, 37 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent ! Depuis plusieurs années, nous entendons la même musique : le gentil Gouvernement d'un côté, prêt à construire des logements abordables, et, de l'autre, les vilains élus locaux qui ne font rien pour aider. Regardons la réalité en face : quelle est votre stratégie de production de logements et d'aménagement du territoire ? Ces deux éléments sont en effet intimement liés : comment répondre au vieillissement de la population, aux séparations, aux divorces et aux coûts toujours plus élevés des logements ?

? Vous aviez tout pour réussir : les Français aiment la pierre et les taux sont incroyablement bas. Pourtant, fiscalité confiscatoire, plafonnement des loyers, protection insuffisante des propriétaires font que les petits investisseurs renoncent à louer ou à contribuer à la production de logements.

ce mandat. Emmanuel Macron faisait part, dès 2017, de son intention de lutter contre la « rente immobilière », considérant même que l'immobilier ne créait pas d'emplois. Vous avez cassé la confiance d'une part des Français et des élus locaux par les menaces permanentes que vous faites planer au-dessus de leur tête.

Nous avons amélioré le bail réel solidaire, lequel permet l'accès à la propriété sans avoir à acheter le foncier, notamment en lui appliquant la TVA à 5,5

saluer. Cela permettra à mon sens d'atteindre l'objectif ambitieux que nous nous fixons en matière de rénovation des passoires thermiques. La stratégie du Gouvernement est donc claire. Elle porte sur la construction comme sur la rénovation.

mais des difficultés apparaissent pour loger la population locale ou héberger certains publics, à commencer par les saisonniers. Dans les territoires de montagne, le marché de l'immobilier est principalement alimenté par les ventes et achats de résidences secondaires, dans certaines communes, représentent plus de 50 % du parc immobilier. Cette situation a pour conséquence une pression à la hausse sur les prix, qui rend plus difficilement accessible la location ou l'achat de biens par et pour les populations locales. La construction de logements sociaux

le conventionnement de loyer social en zone tendue. Si ce mécanisme a du sens, le taux de décote est trop important, particulièrement pour les logements conventionnés situés en zone C.

Aussi, madame la ministre, quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour faire face à cette situation et permettre de transformer des logements vacants en logements sociaux et en logements d'habitation pérenne ? La

à louer leurs biens à loyer maîtrisé. Cela permet de créer du logement abordable dans le parc privé existant. C'est donc un outil précieux dans la lutte contre les vacances de logement.

pour un conventionnement social que pour un conventionnement intermédiaire. La réduction sur les revenus fonciers sera remplacée par une réduction d'impôt proportionnelle aux loyers perçus par les bailleurs, ce qui permettra de toucher davantage de propriétaires. Enfin, les nouvelles conventions du dispositif « Louer abordable » pourront être signées à partir du 1 avril

dite Climat et résilience, entend intensifier la lutte contre l'artificialisation des sols. Elle fixe des objectifs ambitieux : zéro artificialisation nette en 2050 et division par deux du rythme de consommation des espaces naturels par rapport à la dernière décennie. Madame la ministre, sur ces travées, personne ne nie l'urgence de préserver la biodiversité ni celle de changer nos politiques de logement pour limiter l'imperméabilisation des sols. Cependant, ne confondons pas vitesse et précipitation. De tels choix doivent être réfléchis et les élus doivent Partout, dans les territoires ruraux, les élus sont inquiets et demandent l'application différenciée de ces objectifs. Une même politique ne peut être appliquée partout de la même façon, au risque de pénaliser les zones rurales. En effet, comment réduire de 50 % les surfaces constructibles, quand on n'a pas, ou peu, construit ces dix dernières années ? Comment maintenir des écoles ouvertes avec l'interdiction de construire pour accueillir de nouvelles familles ? La ruralité connaît un regain d'attractivité avec la crise sanitaire.

Maintenant que le constat est dressé, madame la ministre, comptez-vous écouter les élus et mettre en place une application différenciée permettant de prendre en contre les particularités rurales ?

qui doit être concilié avec nos impératifs de transition écologique. Les communes rurales représentent environ 14 % de la consommation d'espace pour 4 % de l'augmentation du nombre de ménages. de ménages. Elles font donc face à des enjeux majeurs d'aménagement du territoire et ont tout intérêt à se doter d'un document d'urbanisme afin d'être pleinement maîtres de leur aménagement et de délivrer leurs permis de construire. Ces communes disposent de plusieurs outils incitatifs en faveur de la construction de logements.

accessible en zone détendue. Restent trois points essentiels concernant la lutte contre l'artificialisation des sols. Premièrement, l'objectif « zéro artificialisation nette » est fixé dans la loi à 2050. Deuxièmement, la loi Climat et résilience prévoit précisément que la division progressive du rythme de l'artificialisation des sols soit territorialisée et adaptée aux réalités locales. Troisièmement, nous avons bien entendu les inquiétudes des territoires ruraux, en particulier s'agissant de la dynamique démographique, car ceux-ci pourraient être pénalisés dans leur capacité à se développer. C'est pourquoi les préfets de département accompagneront les communes rurales qui le souhaitent dans l'expression de leur besoin de consommation d'espace.

de disposer d'un accès à internet fiable. Conjuguée à la pénurie de l'offre, cette augmentation de la demande accentue une tension déjà présente. Mon département, l'Oise, connaît, en outre, une croissance démographique plus importante qu'à l'échelle nationale. La situation des jeunes, qui souhaitent accéder à la propriété, mais aussi celle des plus fragiles, est particulièrement préoccupante, alors que le pouvoir d'achat de ces publics est souvent plus faible que dans les zones urbaines. Or, quoi que l'on ait pu entendre, la maison individuelle reste dans nos territoires, en dehors de la capitale et de sa proche banlieue, la norme et un objectif à mon sens légitime. Des dispositifs bienvenus ont été mis en place pour la rénovation dans l'ancien ou pour les centres-bourgs, ces villes dont les centres se sont vidés ces quarante dernières années. Dans certaines d'entre elles, la douceur de vivre a endormi l'acuité visuelle et l'indolence a trop fait oublier l'essentiel : il n'y a pas d'immobilier sans vie. vie. La politique en la matière reste pourtant encore trop concentrée sur la ville. Il vous faut regarder plus loin, car on ne parviendra jamais à loger tous les ménages dans les métropoles de notre pays, à plus forte raison alors que les aspirations de nos compatriotes évoluent vers un certain retour à la nature. Les deux facettes territoriales de la France méritent, l'une comme

pour les communes, de se doter de documents d'urbanisme afin de maîtriser l'urbanisation sur leur territoire et de délivrer des permis de construire. La très grande majorité de nos communes, y compris rurales, sont compétentes en la matière et ont élaboré un document d'urbanisme.

c'est le préfet qui instruit et délivre les permis de construire, mais uniquement en zone urbanisée. Pour toutes les communes dotées d'un document d'urbanisme, les permis de construire sont à la main

avoir une population faible n'est pas un frein pour se doter d'un tel outil ; il est faux de penser que les communes rurales n'ont pas de solution à leur disposition pour construire des logements. Les documents d'urbanisme sont la clé et

sommes aussi dans un beau département, qu'il convient de protéger ; le réseau Natura 2000 nous oblige. Enfin, comme nous sommes dans un département agréable, le télétravail s'y est largement développé au cours de ces deux dernières années. Nos terrains sont de plus en plus prisés et leurs prix augmentent

toujours aussi hors sol- voire hors hémicycle, comme c'était le cas hier soir ! Madame la ministre, les problématiques que rencontrent ces communes ne sont pas de gauche ou de droite : elles sont factuelles et il faudra leur apporter une réponse. En somme, ne pensez-vous pas qu'il serait tout de même utile, afin de vous éviter de vous prononcer sur chaque commune de France, de faire enfin confiance, au moins, à vos préfets afin d'adapter nos ambitions à la réalité des territoires ? La parole est à Mme la ministre

triennaux 2017-2019 et seulement 280 sont carencées. Cela démontre donc cette bonne foi des élus. C'est précisément en tenant compte de ce bilan et de l'impératif de continuer à construire des logements sociaux dans les territoires qui en manquent, tout en prenant en compte les contraintes locales, que le Gouvernement a proposé la pérennisation et l'adaptation du dispositif SRU dans le projet de loi 3DS. Il a ainsi supprimé la date butoir de 2025 de 2025 et fixé un taux de rattrapage par période triennale de 33 % du déficit, ce qui est réaliste et atteignable. Enfin, il a créé des contrats de mixité sociale (CMS) signés par le préfet, la commune et l'intercommunalité, afin de déterminer les moyens et les modalités de déploiement de la trajectoire de rattrapage de la commune. Ces contrats peuvent prévoir, durant deux périodes triennales au maximum, un taux dérogatoire de rattrapage du déficit limite pour tenir compte des spécificités et des contraintes locales que vous avez évoquées. L'examen parlementaire a permis de procéder à un certain nombre d'ajustements, en particulier de recourir à un CMS fixant un taux de rattrapage dérogatoire sans limite de durée pour les communes ayant une part importante de leur territoire grevée d'inconstructibilité, ainsi que pour les communes de moins de 5 000 habitants. Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, nous agissons en responsabilité en tenant compte des spécificités des territoires, tout en répondant à l'impératif de construction de logements.

Dans la commune du Bignon, située dans le vignoble nantais, le prix du foncier a augmenté de 67 % en quatre ans. À Saint-Père-en-Retz, dans le pays de Retz, le prix des terrains a été multiplié par trois ces deux dernières années.

à des injonctions contradictoires qui deviennent impossibles à tenir. Ils voient arriver dans leur commune des ménages aux revenus confortables, tandis que les jeunes quittent leur territoire. Madame la ministre, ma question est simple pourquoi avoir voulu imposer par le haut ce zéro artificialisation nette ? Comment entendez-vous faire appliquer cette loi de la même manière dans un département qui perd des habitants et dans un département qui en gagne 17 000 chaque année ?

déjà répondu sur la question du foncier, je reviendrai sur celle de l'artificialisation des sols. Permettez-moi de vous redonner quelques chiffres : aujourd'hui, 3,5 millions d'hectares sont artificialisés en France. Ramené à la population, c'est 15 % de plus qu'en Allemagne

madame la sénatrice -, nous avons inscrit dans la loi la prise en compte des efforts déjà réalisés par les territoires. Enfin, pour répondre aux inquiétudes des associations de collectivités, nous avons introduit dans le projet de loi 3DS un allongement

En effet, ces territoires se trouvent dans des situations critiques en matière de logement en raison de leur proximité avec des pays plus riches, où les salaires sont plus élevés. C'est en particulier le cas des départements qui se trouvent à côté de la Suisse et du Luxembourg. Cette proximité entraîne une hausse des loyers très importante. De ce fait, les personnes qui ne travaillent pas dans un pays frontalier rencontrent de très grandes difficultés à trouver des logements à des prix abordables. Cette hausse des prix des logements entraîne des difficultés de recrutement pour les entreprises, mais aussi et surtout dans les services publics. En effet, les fonctionnaires ne souhaitent plus s'installer dans ces régions, car ils savent qu'ils ne pourront pas y vivre dignement du fait des loyers exorbitants. Tous les professionnels sont touchés : saisonniers, agents administratifs, personnels de santé, policiers et j'en passe. La situation commence à devenir critique et il est de notre devoir de trouver des solutions.

entreprises, dit Pinel, ayant pris fin au 1 janvier, il peut être envisagé de mettre en place un dispositif similaire prévoyant des crédits d'impôt en contrepartie d'un engagement à louer à prix modéré dans les zones frontalières où la situation du logement est tendue.

avec les marchés locaux et une égalité de traitement de l'ensemble des propriétaires. De plus, ce dispositif a été transformé en une réduction d'impôt dont le taux est directement lié à l'effort de loyer consenti par le propriétaire. Concernant l'éligibilité au dispositif Pinel et le zonage,

à ce département, encore une fois afin de tenir compte des particularités locales. Le ministère du logement travaille en lien avec Bercy et le préfet pour définir la liste

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, un chiffre donnera la mesure de la crise du logement que connaît notre pays : selon l'OCDE,

par la mission Girometti-Leclercq au mois de septembre dernier. Dans le même temps, les inégalités entre les territoires persistent. Jean-Louis Borloo l'a souligné dans un rapport qui a connu un retentissement important, mais qui n'a guère été pris en compte par ce gouvernement, qui l'avait pourtant commandé : sur les 1 500 quartiers politique de la ville, 216 connaissent des difficultés urbaines, 60 sont en risque de fracture et 15 en risque de rupture, de sorte que 10 millions de nos concitoyens se considèrent comme relégués. La difficulté de nos concitoyens à trouver un logement se répercute jusqu'à l'hébergement d'urgence : 200 000 personnes sont hébergées dans des structures d'urgence, plus de 70 000 l'étant dans des hôtels. L'ensemble de la chaîne de la politique du logement paraît bloqué

Le Gouvernement a annoncé l'agrément de 250 000 logements sociaux en deux ans, mais cet objectif ne sera clairement pas atteint, et le déficit de l'année 2020 ne sera probablement pas rattrapé. Un élément parmi d'autres : la hausse annoncée du taux du livret A au 1 février 2022 renchérit mécaniquement le coût des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux bailleurs sociaux et pèsera nécessairement sur le modèle de financement des projets sans pour autant rendre le livret A véritablement intéressant pour les épargnants modestes en raison du niveau de l'inflation. Loin du choc d'offre annoncé, la politique du logement semble s'être concentrée sur la promotion de la rénovation des logements, qui est, elle, en forte croissance. Si cette politique doit être approuvée dans ses objectifs, car elle est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques, elle ne répond pas au besoin fondamental de logement qui est de plus en plus difficile à satisfaire dans notre pays. Or les cinq années passées ont surtout été marquées par la recherche d'économies : la contribution de l'État au financement des APL est passée de 15,5 milliards d'euros en 2007 à 13 milliards d'euros en 2022, tandis que le cofinancement assuré par les employeurs demeurait stable. APL consacrées à l'accession à la propriété ont été supprimées, alors qu'elles jouaient un rôle important dans l'acquisition de logement par des ménages modestes. Les locataires ont vu leurs APL diminuer de 5 euros en 2017, tandis que les bailleurs ont, pour leur part, été contraints de rogner sur les frais d'entretien ou d'investissement du fait de la mise en place de la réduction de loyer de solidarité (RLS). Cette année, c'est le versement contemporain des aides qui, après plusieurs années de retard et quelques dysfonctionnements, a été mis en place. L'État s'est ainsi désengagé en partie du soutien au logement des Français modestes, de même qu'il a cessé ses contributions budgétaires au financement des logements sociaux au travers du Fonds national des aides à la pierre (FNAP). L'État se repose donc sur les bailleurs sociaux et sur des acteurs tiers, notamment Action Logement qui a régulièrement été appelé à contribuer au financement des principaux dispositifs de la politique du logement et de la ville. Or les marges financières de cet organisme sont désormais largement entamées, et la question du financement des aides à la pierre par exemple, être posée, si Action Logement n'apporte plus 350 millions d'euros au FNAP à partir de 2023. Tout en réduisant les financements, l'État accroît les contraintes pesant sur l'ensemble des acteurs le coût de l'ensemble des réglementations, notamment thermiques, est de plus en plus élevé pour les acteurs du bâtiment, qui sont également soumis à la hausse des coûts de l'énergie et à une crise d'approvisionnement de certains matériaux.

Les collectivités locales sont soumises à des injonctions difficiles à concilier : accroître la production de logements de qualité pour la population, notamment afin de remplir les critères de la loi SRU, et favoriser le développement économique local, mais sans utiliser plus de terrain qu'aujourd'hui. contrairement à la rénovation énergétique, la lutte contre l'artificialisation ne s'accompagne que d'un faible soutien : l'action de l'État passe essentiellement par la fixation de normes que d'autres, au premier rang desquels les collectivités, devront appliquer. Comme l'a démontré le succès du fonds pour le recyclage des friches qui a dû être doublé, les besoins sont importants et les collectivités ne manquent pas de projets. Toutefois, ce fonds n'épuise pas le sujet, tant s'en faut. L'État doit mieux accompagner les collectivités face à ces défis, par exemple pour la révision de leurs documents d'urbanisme. Trois grands axes devront donc être posés : la production de logements nouveaux, l'amélioration de la performance énergétique du stock de logements et l'annulation progressive de toute artificialisation nouvelle des sols. Ces trois objectifs sont dispersés au travers d'un ensemble de mesures de toute nature reposant à la fois sur l'État, les collectivités et les acteurs privés.

Comment accepter que de l'argent public soit donné à des États qui, en parallèle, n'acceptent pas une convention avec la France sur la réintégration ?

Il me semble important, dans le cadre de ce propos liminaire, de revenir sur le contexte migratoire dans lequel ce texte important a été déposé par le Gouvernement et adopté par le Parlement. Ce contexte est bien sûr celui de l'après-crise migratoire de 2015-2016, dont chacun se souvient. La France restait alors exposée à une forte pression migratoire à ses frontières nationales, comme en témoigne le nombre des non-admissions d'étrangers en situation irrégulière à nos frontières-

121 200 demandes d'asile, dont 36 % de demandeurs d'asile dits Dublin, c'est-à-dire ayant déposé une première demande dans un autre pays de l'Union européenne.

Le débat au Parlement a permis d'enrichir le projet du Gouvernement dans le parfait respect de notre Constitution, puisque, fait inédit pour une loi relative à la question de l'immigration, le texte a été validé dans toutes ses dispositions par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 septembre 2018. Il a donc pu entrer en vigueur de manière progressive entre le 11 septembre 2018 et le 1 mars 2019, le temps de prendre les quarante mesures réglementaires requises pour son application effective. J'en viens à présent à l'atteinte des objectifs fixés par la loi, puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. En matière d'asile, l'objectif principal était de pouvoir traiter la demande dans un délai de 6 mois, recours contentieux compris. Nous progressons dans cette voie. Le délai moyen d'enregistrement en préfecture est maîtrisé depuis fin 2020, puisqu'il est de 2,7 jours, et ce grâce au travail de renforcement des guichets uniques pour demandeurs d'asile, qui regroupent les effectifs des préfectures

Je souligne toutefois que la productivité mensuelle de l'Ofpra a progressé d'environ 25 % grâce à l'effet combiné des mesures d'organisation et des renforts en effectifs. En effet, nous avons souhaité financer plus de 200 équivalents temps pour atteindre le nombre d'environ 12 000 décisions mensuelles au mois de septembre 2021. L'Ofpra a donc adopté plus de 127 000 décisions cette année. Cela correspond à un pic d'activité jamais atteint, qui en fait le premier office de protection au sein de l'Union européenne en termes de niveau d'activité devant l'Allemagne. Je salue d'ailleurs le travail délicat et parfois éprouvant mené par les agents de l'Ofpra. La baisse du « stock de dossiers » en cours d'instruction témoigne elle aussi de cette activité soutenue, puisque ce stock est passé de près de 88 000 dossiers au mois d'octobre 2020 à 50 000

de 2018 prévoyait également le principe de l'orientation directive des demandeurs d'asile, laquelle a été mise en oeuvre le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés (Snadar) 2021-2023. Entré en vigueur le 1 janvier 2021, il prévoit de rééquilibrer la prise en charge des demandeurs d'asile sur le territoire en desserrant la capacité d'accueil francilienne au profit de régions qui sont moins tendues à cet égard.

Ce dispositif s'appuie sur le renforcement de la capacité du parc d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile. Grâce à la création de près de 4 700 places en 2021, le dispositif comporte environ 103 000 places

AEM n'étant pas obligatoire à ce jour, celui-ci a été utilisé au 1 juillet 2021 par 78 collectivités. Pour favoriser le déploiement de l'outil sur l'ensemble du territoire national, un mécanisme d'incitation financière est opérant depuis le 1 janvier 2021 d'août 2021, sur 19 441 dossiers enregistrés, 95 % des personnes déclarées comme MNA sont des hommes. Les majeurs représentent plus de 50 % des décisions prises par les présidents de conseils départementaux. La répartition par nationalité et stable

est d'attirer davantage d'étrangers très qualifiés et de mieux les accueillir. À cette fin, la loi a ouvert de nouveaux cas de délivrance du passeport talent. Je pense aux entreprises innovantes souhaitant recruter des étrangers non diplômés en France : la loi a ainsi assuré la transposition de la directive concernant

enfin, nous allons rétablir nos frontières ! Enfin, nous allons punir ces millions de fraudeurs à la carte Vitale et aux prestations sociales ! Enfin, nous allons expulser les clandestins et les criminels étrangers de manière définitive parliez non pas des étrangers, mais des Français, ces Gaulois réfractaires non vaccinés. Contre eux, vous êtes prêts à violer tous les principes de notre État de droit. Nous n'oublierons pas Nous n'oublierons pas que l'État de droit devient accessoire, quand il s'agit de protéger des vies humaines, puisque c'est ainsi que vous justifiez vos mesures liberticides. Nous saurons nous en rappeler quand nous abrogerons le regroupement familial : si l'on peut suspendre la liberté de circuler pour les Français, il n'y aura donc aucun problème à le faire pour les étrangers ! Nous saurons nous en rappeler quand nous équiperons les immigrés d'une application de afin de pouvoir vérifier qu'ils quittent bien le territoire à l'expiration de leur titre de séjour. rien changé : le nombre de titres de séjour a explosé en 2019, avec 277 000 délivrances, dont 14 % seulement concernait une immigration de travail. Cette immigration économique est non pas une chance, mais un fardeau. Du point de vue sécuritaire et identitaire, elle est un fléau. N'oublions pas les clandestins. Dans cet hémicycle,

vous préfériez les répartir chez nous. Il a même estimé qu'il y allait de « l'honneur de la France ». Alors que 115 000 demandes d'asile ont été rejetées en 2019, seules 19 000 expulsions forcées ont eu lieu. Cela fait donc 95 000 clandestins supplémentaires sur notre sol, soit l'équivalent d'une ville comme Tourcoing. Madame la ministre, ma question est la suivante

En France, la proportion d'immigrés dans notre population se situe dans la moyenne de l'Union européenne : hormis l'Italie, tous nos voisins proches connaissent des proportions d'immigrés bien supérieures.

Madame la ministre, pourquoi ne dénoncez-vous pas les propositions relatives aux quotas, totalement irresponsables, dans la mesure où nous n'avons pas de marge de manoeuvre, puisque nous délivrons peu de titres de séjour tous les ans ? Pourtant, 220 000 titres

l'examen de ce texte, s'élevaient encore en moyenne à onze mois. À cette fin, la loi a doté les acteurs de nouveaux outils, s'agissant notamment des modalités de convocation et d'entretien, ou encore de déclenchement de la procédure accélérée, afin que la question de la régularité du séjour soit tranchée avec diligence.

et pour cause : le droit d'asile est massivement détourné par des migrants qui désirent s'établir en France. Or force est de constater que la majorité d'entre eux ne relèvent pas du droit d'asile. Les protections offertes par cette procédure, que nous devons garantir, mais aussi encadrer, en font un canal privilégié d'immigration.

qu'à condition que les accords conclus avec les pays tiers concernés comportent des garanties solides, notamment en matière de respect des droits fondamentaux. Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le Président de la République a annoncé son souhait de faire avancer le pacte migratoire. Cela permettra, d'une part, de mieux harmoniser les règles en matière d'asile entre les pays européens, en particulier

oui ! Certes, il est d'une évidence implacable que ce défi de civilisation ne peut pas être relevé en quelques semaines, simplement par l'adoption d'une loi. Néanmoins, la question de l'effectivité de la loi Asile et immigration par rapport aux objectifs initiaux affichés se pose très sérieusement.

Ce taux d'exécution interroge sur la crédibilité de nos institutions et révèle un certain manque de volonté politique du Gouvernement, malgré sa communication abondante dans ce domaine.

Ce chiffre, couplé au taux d'exécution des OQTF, laisse imaginer le nombre de personnes demeurant illégalement sur notre territoire. Madame la ministre, face à cette triste réalité, ne serait-il pas temps de traiter les demandes d'asile à l'extérieur des frontières européennes, par exemple dans les ambassades et les consulats des États membres de l'Union européenne situés dans les pays d'origine ? Cela permettrait un traitement local plus rapide des demandes d'asile légitimes au bénéfice des demandeurs se trouvant parfois dans des situations dramatiques et dont l'accueil et la protection honorent la France. Madame la ministre, est-ce une mesure que le Gouvernement auquel vous appartenez compte proposer à l'échelon européen afin de renforcer notre réponse en matière d'asile et notre arsenal en matière migratoire ? La parole est à Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur, un dispositif de traitement des demandes d'asile dans les pays tiers à l'Union européenne soulève à ce stade de très- trop ! - nombreuses interrogations. Celui-ci serait peu opérationnel, parce qu'il impliquerait un accord des pays tiers concernés

en dehors du territoire de l'Union européenne, notamment au Proche-Orient ou en Afrique. Il nous semble par ailleurs assez peu réaliste de penser que cela puisse mettre fin à la migration de demandeurs d'asile vers le territoire européen. Du point de vue juridique, si ce dispositif devait remplacer le système actuel de demandes d'asile sur le sol français, il entrerait en contradiction avec un certain nombre de principes fondamentaux inscrits dans notre Constitution, ainsi qu'avec nos engagements européens. En revanche, il est vrai que la recherche d'un système de l'asile plus efficace justifie de consolider le dispositif de recueil des demandes d'asile à la frontière extérieure de l'Union européenne. Cette orientation, figurant au coeur du pacte sur la migration et l'asile proposé par la Commission européenne, est soutenue par la France.

l'immigration est un phénomène naturel, lié à des contextes climatique, socio-économique, humanitaire et géopolitique. La question devrait être la suivante : comment recevoir en France des immigrés de façon humaine et acceptable socialement afin de permettre une intégration réussie, à l'image de celles et de ceux ayant contribué à la richesse de notre pays La maîtrise de l'immigration doit s'entendre, non pas comme une limitation quantitative dont je peine à voir, à moins de tomber dans l'arbitraire, quels pourraient être les critères concrets et légaux, mais comme l'accompagnement de ce phénomène naturel.

quotas annuels ? Souhaite-t-il instaurer une immigration choisie en fonction des compétences, de la politique étrangère de la France ou d'autres critères bien moins catholiques ? Que faire après avoir reçu et mal traité ces nouveaux arrivants ?

que ses moyens sont administrés par le Conseil d'État. En tout état de cause, la CNDA constitue un acteur essentiel de la chaîne de l'asile. Le renforcement de ses moyens et de sa capacité décisionnelle est déterminant pour que l'objectif d'un délai moyen de procédure soit ramené à 6 mois.

Pour ma part, je me concentrerai sur le niveau réel d'atteintes portées à nos valeurs fondamentales depuis trois ans, qu'il s'agisse du respect du droit d'asile ou, tout simplement et plus généralement, du respect de la dignité de la personne humaine.

en réalité, fait le tri entre les enfants à protéger et ceux qu'il faut encore davantage fragiliser, tels que les mineurs non accompagnés. Les présidents des conseils départementaux sont aujourd'hui contraints d'utiliser ces fichiers et de solliciter le concours du préfet. Cette logique répressive et de défiance grandissante à l'égard de ces enfants en grande précarité et vulnérabilité doit être définitivement renversée. Elle doit cesser. Le sujet

les migrants en rétention administrative le temps de la pandémie. Au contraire, environ 28 000 personnes y ont été enfermées en 2020, et guère moins depuis, malgré la situation sanitaire. Certaines d'entre elles souffrent de pathologies lourdes, mettant en lumière l'absence d'accès effectif aux soins en rétention. Ma question est simple

Avant cet événement dramatique, l'évacuation d'un camp, dimanche dernier, avait été précédée d'affrontements entre des migrants et des membres des forces de l'ordre. Des policiers avaient alors été blessés. Sans qu'il faille établir un lien entre ces deux événements, l'on constate que ce territoire est en proie à une situation qui, malheureusement, s'enlise chaque jour un peu plus dans la violence et la misère. Bien sûr, chacun le déplore. Force est de constater que la loi Asile et immigration ne semble pas avoir permis de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les Calaisiens depuis des années. Indépendamment, là encore, des gouvernements successifs, c'est une réalité qui s'impose à nous. Rappelons que la fermeture du centre de Sangatte date du mois de décembre 2002- voilà dix-neuf ans maintenant -et le démantèlement de la première jungle de Calais de 2009.

témoigné votre soutien aux forces de l'ordre et à l'ensemble des élus- à commencer par Natacha Bouchart -qui sont mobilisés aux côtés de l'État. Cela étant, nous souhaitons vraiment des avancées dans la coopération avec la Grande-Bretagne.

loi sur l'immigration et l'asile depuis 1980, elle n'est pas la première à avoir tenté d'assurer un accueil des migrants dans la dignité. Cependant, des campements de fortune continuent de s'établir sur notre territoire. Ils ne peuvent évidemment pas garantir à leurs occupants les conditions de sécurité et de salubrité les plus élémentaires. On l'a vu dans mon département, à Lyon, dans les quartiers des pentes de la Croix-Rousse ou encore de la Confluence : on peine à trouver à chacun des solutions d'hébergement de long terme, certains migrants se tournant alors vers des squats. La question de la répartition des arrivants sur le territoire est au centre de cette problématique. Lyon, en particulier, constitue une terre d'accueil significative. Ainsi, 28 % des demandes d'asile effectuées en région Auvergne-Rhône-Alpes sont déposées à Lyon. D'ailleurs, la région est la deuxième la plus sollicitée en termes de nombre de demandes. Deuxième plus sollicitée, elle n'est cependant que la quatrième au classement du nombre de centres d'accueil et d'orientation après l'Occitanie, le Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine. En effet, la question de l'orientation des migrants est indissociable de celle du caractère suffisant des infrastructures d'accueil. La loi Asile et immigration, en son article 13, traitait pourtant de ces questions, avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés. Elle prévoit que celui-ci fixe la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région, ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. Madame la ministre, face aux conditions d'accueil insatisfaisantes dont nous sommes témoins, ne faut-il pas revoir les dispositions de la loi concernant l'hébergement ?

ont été réalisés, notamment grâce à la mise en oeuvre des dispositions votées par le Parlement dans la loi de 2018. Les capacités au sein du dispositif national d'accueil, par exemple, ont été considérablement renforcées. En 2020, 4 500 nouvelles places ont été financées ; elles sont aujourd'hui ouvertes en quasi-totalité. Par ailleurs, on compte 400 places supplémentaires dédiées aux réfugiés vulnérables en Île-de-France et 6 000 nouvelles places pour les demandeurs d'asile et les réfugiés.

d'orientation des demandeurs d'asile depuis les régions les plus tendues, en particulier l'Île-de-France, sont effectives depuis le début de l'année 2021, comme je le précisais dans mon propos liminaire. En un an, ce dispositif a permis d'orienter plus de 15 000 demandeurs d'asile vers un hébergement

afin de dénoncer l'augmentation du nombre de décisions rendues par ordonnance, c'est-à-dire sans que le demandeur soit entendu lors d'une audience. Les agents de la CNDA, ainsi que les avocats, ont dénoncé à cette occasion une « politique du chiffre ».

-que les délais d'examen des demandes soient réduits. Pour autant, il n'est pas justifié que des personnes en situation très difficile, venant de pays sûrs ou non, ayant subi des persécutions, notamment dans les pays dits non sûrs, ne puissent faire valoir leurs droits oralement, s'expliquer,

mais dans le respect des droits des demandeurs d'asile à être entendus avant qu'une décision ne leur soit signifiée ? La parole est à Mme la ministre

de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si la crise sanitaire a conduit, en 2020, à un allongement conjoncturel des délais de traitement des demandes, la situation a connu une amélioration sensible depuis la fin de l'année.

Nous qui sommes au contact de la réalité constatons chaque jour les ravages de l'ensauvagement, notamment lié à l'immigration. Il est vrai qu'en ce domaine M. Darmanin avait de prestigieux prédécesseurs ... Je me souviens, ici même, de M. Manuel Valls défendant solennellement que l'on trie parmi les réfugiés. Les morts du Bataclan ont payé cet angélisme ! Au terme de ce quinquennat, je souhaite savoir comment le ministre de l'intérieur juge la situation actuelle de la politique migratoire, de la lutte contre l'immigration clandestine, de l'immigration légale et de l'intégration. Je constate que l'immigration clandestine n'a jamais autant prospéré. Le ministre lui-même parle de 600 000 à 700 000 clandestins présents sur notre sol. Pourtant, M. Emmanuel Macron, au début de son quinquennat, promettait d'expulser 100 % des clandestins. Paroles, paroles ... Quant à l'immigration légale, elle est largement liée au regroupement familial, donc non choisie. Or le regroupement familial a été adopté sous réserve que l'immigré ait les moyens de faire vivre sa famille. Quand on sait que le taux de chômage des immigrés extra-européens atteint 24 %, on peut douter que cette immigration légale soit conforme à l'intention du législateur ! De plus, combien d'immigrés légaux viennent grossir les rangs de l'immigration clandestine après l'expiration de leur visa ? Nous délivrons 3,5 millions de visas à l'année ! En d'autres termes, que fait-on pour que l'immigration légale soit réellement une immigration choisie ? En cinq ans, nous avons entendu beaucoup de discours, mais les problèmes ont empiré. Je ne rappellerai pas ici les propos du ministre de l'intérieur Quand saurons-nous enfin ne serait-ce que le coût de l'immigration ? Trouvez-vous raisonnable, madame la ministre, alors que les Français ont des difficultés à se loger et à se soigner, d'accueillir près de 450 000 personnes tous les ans ?

Une loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ... Comme c'est souvent le cas, l'intitulé de la loi du 10 septembre 2018 pourrait donner l'impression que, ça y est, le Parlement a adopté la réforme permettant de régler les questions liées tant à l'immigration qu'à l'intégration. ans après, ce texte n'a pas atteint ses objectifs- disons, pas encore. Sans trop vouloir réduire le champ de notre débat, un sujet que nous avons à traiter en la matière est, bien évidemment, l'éloignement de tous les étrangers sans droit ni titre présents sur le territoire national. Le texte de 2018 visait à raccourcir les délais de traitement des demandes, notamment d'asile, objectif que nous avons naturellement toujours partagé. s'assurer de l'exécution des obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, c'est mieux ! Après s'être élevé jusqu'à 22 % en 2012, le taux d'exécution des OQTF a connu une forte baisse, ne dépassant plus plus 15 % depuis 2016 et se situant même en dessous de 13 % en 2018, comme en 2019. Son niveau a atteint des planchers très bas avec la crise du covid. Ce n'est pas un reproche fait à la ministre présente mais cela interroge néanmoins sur la crédibilité du discours de la France. Au-delà des améliorations techniques prévues par le texte de 2018, le coeur du problème reste aujourd'hui celui-là. C'est d'ailleurs une question au moins autant de volonté politique que d'innovation législative.

Les éloignements contraints atteignent ainsi un niveau inédit en 2019, avec 20 994 mesures exécutées, soit une augmentation de 34 % par rapport au niveau de l'année 2016, pour ne prendre que cet exemple. Cette dynamique, chacun le sait, a été interrompue par la crise sanitaire et la fermeture des frontières, ayant entraîné

c'est-à-dire essentiellement sortant de prison, radicalisés, représentant une menace. Les moyens de notre dispositif d'éloignement ont été accrus. Le nombre de places de rétention sera porté en métropole à 2 200 à l'horizon de 2024,

places seront financées dans le cadre du plan France Relance. Enfin, la fermeté du ministre de l'intérieur, qui a sensiblement réduit la délivrance des visas au profit des pays les plus récalcitrants à délivrer des laissez-passer consulaires, est une preuve supplémentaire de l'engagement ferme et concret du Gouvernement pour obtenir une meilleure exécution des OQTF. La parole

l'augmentation moyenne de la proportion des personnes nées à l'étranger est passée de 11,6 % en 2010 à 13,1 % en 2020, soit 1,5 point d'augmentation. Au sein de l'OCDE, la moyenne s'est établie à 2,2 points sur la décennie.

On peut alors imaginer que c'est le taux d'exécution des OQTF qui préoccupe certains d'entre vous, mes chers collègues. Cela n'est d'ailleurs pas la première fois que l'on se focalise plus que de raison sur ce sujet, qui se révèle souvent périlleux. M. Macron, lui-même, a dans, au mois d'octobre 2019, affirmé son engagement de faire procéder à 100 % des OQTF d'ici à la fin de son mandat. Il est évidemment difficile d'accepter que des décisions de l'administration française ne soient pas appliquées. On connaît un obstacle évident à cette bonne application : la France est tributaire des laissez-passer délivrés par les pays tiers. Il y a cependant un autre obstacle, qui se situe sur notre territoire : il se trouve que l'on délivre des OQTF à des personnes n'ayant pas lieu d'être éloignées

avant de débattre de taux, de chiffres, de statistiques, regardons déjà ceux à qui l'on impose ces OQTF. Certains, parce qu'ils causent des troubles à l'ordre public, doivent être éloignés, mais ils n'ont rien à voir avec ces étrangers intégrés, notamment les jeunes majeurs, que l'on s'acharne à vouloir éloigner sans raison légitime.

d'abord, la voie de plein droit pour les mineurs isolés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, au plus tard à l'âge de 16 ans. Cette voie a fait ses preuves. Il y a, ensuite, une voie d'admission exceptionnelle au séjour pour ceux qui sont pris en charge entre 16 et 18 ans, et qui justifient d'au moins six mois de formation professionnelle sous certaines conditions. C'est exactement la situation que vous avez décrite, monsieur le sénateur. La circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls, sur l'admission exceptionnelle au séjour permet par ailleurs de traiter certaines situations particulières n'entrant pas dans ce cadre,

chers collègues, le bilan que nous pouvons en faire est accablant. Madame la ministre, je tiens à partager avec vous trois constats, montrant à quel point la situation est grave. D'abord, vous avez délivré plus de 275 000 titres de séjour en 2019. C'est 20 % de plus en trois ans. Je rappellerai que vous avez même étendu la réunification familiale aux frères et soeurs des réfugiés mineurs. Par ailleurs, 31 188 admissions exceptionnelles au séjour ont été enregistrées en 2019, soit 63 % de plus que sous le mandat de Nicolas Sarkozy.

Non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais elle s'est fortement détériorée. Mon collègue Sébastien Meurant propose depuis de longs mois la création d'une mission d'information sur le coût de l'immigration. Ma question est simple, à combien estimez-vous le coût global réel de l'immigration pour la France ? Allez-vous enfin lever ce tabou ? Bravo ! La parole est est à Mme la ministre déléguée. En matière de politique d'immigration et d'intégration, le budget de l'État fait l'objet chaque année d'un document de politique transversale, qui est adossé au projet de loi de finances.

pour l'année 2021. Cette somme englobe, à la fois, des dépenses engagées directement au titre de la politique publique d'immigration, d'asile et d'intégration des primo-arrivants, les coûts engagés par les forces de sécurité pour lutter contre l'immigration irrégulière, mais aussi les dépenses supportées par les ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou des solidarités et de la santé, par exemple au titre de l'aide médicale d'État (AME)- c'est bien normal ! Une approche plus globale suppose de mettre en rapport les coûts

Madame la ministre, à quatre mois de la fin de ce quinquennat, il n'y a plus rien à attendre de votre gouvernement. Ce que vous n'avez pas fait en cinq ans, vous ne le ferez jamais, car vous êtes complaisants et laxistes vis-à-vis d'une immigration que vous voyez, à tort, comme une chance pour la France. Sachez, madame la ministre, que l'immigration illégale et incontrôlée est vécue comme un fardeau de plus en plus pesant par

recoupement des fichiers des titres de séjour, de l'aide médicale d'État ou de la caisse d'allocations familiales. Pourtant, tout se passe comme si personne ne voulait savoir, de peur que cette réalité ne soit gênante pour les pouvoirs publics.

en 2020, Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'immigration, estimait à 900 000 le nombre d'étrangers qui séjournaient illégalement sur le territoire. Malgré l'aveuglement de certains démographes sur cette question, ce chiffre est objectivement inquiétant la France accueille de plus en plus de ressortissants étrangers en dehors de tout canal officiel, alors que nos capacités d'accueil sont de plus en plus saturées et que nos dépenses sociales explosent. Madame la ministre, le Gouvernement doit disposer de données fiables pour bien gouverner et maîtriser l'immigration. Que les Français y aient accès Pouvez-vous nous dire si l'État a fait des progrès dans ce domaine et, surtout, quelle est l'ampleur réelle de l'immigration irrégulière ?

permet une première approche, puisque ce dispositif offre à certains étrangers en situation irrégulière un accès aux soins sous condition de résidence stable, c'est-à-dire avec trois mois de résidence ininterrompue en France. Au 30 septembre 2020, d'après les derniers chiffres dont nous disposons, il y aurait environ 368 890 personnes bénéficiaires de l'AME. À compter de 2022, la mise en place du système européen d'entrée et de sortie devrait permettre d'enregistrer des données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures à l'Union européenne. En l'état, l'activité d'interpellations aux frontières nous donne seulement une indication de la pression migratoire à nos frontières. La parole

Ce système permettrait justement de limiter le nombre d'illégaux et de mesurer plus précisément la réalité de l'immigration. La

Cette disposition, introduite par le Sénat, était très attendue, notamment par les conseils départementaux, qui assurent la prise en charge de ces publics, tant les fraudes et les difficultés sont nombreuses.

Or, trois ans plus tard, force est de constater que les problèmes demeurent, voire s'aggravent. Je n'ai d'ailleurs pas manqué d'interroger le Gouvernement à plusieurs reprises à ce sujet, en particulier après des actes de violences répétées commises par ces personnes autour des gares de mon département. département. Voilà quelques jours, une bagarre au couteau a éclaté entre deux MNA devant le foyer qui les hébergeait à Beauvais. Je rappelle que la politique migratoire relève de l'État, et non des collectivités territoriales. Pourtant, celles-ci continuent d'en assumer les conséquences, y compris financières, avec un impact lourd sur leur budget. Des ajustements législatifs inscrits dans le projet de loi relatif à la protection des enfants sont en cours d'adoption, prévoyant notamment une répartition plus juste des mineurs non accompagnés sur le territoire et la généralisation du recours au fichier national d'appui à l'évaluation de la minorité.

Madame la ministre, allez-vous faire de la gestion des MNA une priorité au sein de votre politique migratoire ?

la protection de l'enfance et pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier d'étrangers en France, dans un contexte d'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés. Ce fichier national permettra non seulement de lutter contre le nomadisme entre départements, mais aussi d'éviter les détournements du dispositif de protection de l'enfance par des majeurs. collectivités, quatre-vingt-deux départements et la métropole de Lyon ont signé une convention avec le préfet territorialement compétent pour l'utilisation de ce fichier, ce qui a permis d'introduire plus de 20 000 dossiers dans cet outil. départements ont décidé de ne pas recourir à ce traitement malgré la création d'un mécanisme d'incitation financière opérationnel depuis le 1 janvier 2021. Or la pleine efficacité du dispositif est conditionnée à sa mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé de rendre obligatoire l'utilisation du fichier AEM sur tout le territoire, disposition insérée dans le projet de loi relatif à la protection des enfants, adopté au Sénat le 15 décembre dernier. La parole

en raison de leur engagement. C'est là le sens premier et la définition de l'asile, c'est-à-dire l'accueil de personnes qui, en raison de leur engagement, sont particulièrement menacées dans leur pays d'origine. Nous avons donc vocation

madame la ministre, mes chers collègues, en 1991, l'ancien Président Valéry Giscard d'Estaing s'interrogeait : « Immigration ou invasion ? » Trente et un ans après, certains pourraient se poser la même question. Aussi, mes chers collègues,

Plus de trois ans après la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, force est de constater que ces problématiques demeurent plus que jamais d'actualité. Certes, on nous dira que les moyens de l'Ofpra et de la Cour nationale du droit d'asile sont en hausse, que la police aux frontières a été mobilisée de manière accrue aux frontières ou que le nombre de places en centre de rétention administrative augmente. C'est éminemment nécessaire, mais cela ne suffit pas, loin de là. là. Les chiffres sont en effet têtus et révèlent le manque de maîtrise des pouvoirs publics sur les flux et les dépenses. Notre collègue Sébastien Meurant l'a bien illustré dans son rapport pour avis du projet de loi de finances pour Il rappelle que le financement de l'allocation pour demandeur d'asile, l'ADA, était en hausse, à environ 467 millions d'euros, mais que ce financement initial avait été quasi systématiquement dépassé lors de l'exécution des budgets précédents. On ne peut donc guère parler de « maîtrise » quand les dépenses excèdent systématiquement les prévisions et qu'une infime fraction seulement de certaines décisions essentielles à l'effectivité de la politique en question fait l'objet d'une exécution ! Cela ne se résume pas à de l'arithmétique. La situation sur le terrain demeure dégradée. Les évacuations de campements sauvages émaillent l'actualité ; notre ancien collègue de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, s'en faisait encore l'écho dans une question d'actualité au Gouvernement il y a un peu plus d'un an. Catherine Belrhiti a également Pendant ce temps, les événements sur les bords de la Manche, à la frontière de la Pologne et en Méditerranée nous rappellent que les flux migratoires se poursuivent et qu'une gestion réaliste et digne de leur accueil s'impose. La baisse temporaire La baisse temporaire de certains indicateurs pendant la durée de la crise sanitaire ne doit pas nous le faire oublier. Face à ce constat, nous ne pouvons plus nous permettre d'hésiter davantage. En raison des évolutions démographiques, géopolitiques et environnementales, la pression migratoire aux frontières de l'Europe ne devrait cesser de croître au cours des prochaines années. Nous le savons, la population africaine devrait doubler d'ici à 2050. Cela impose de renouveler notre droit en profondeur. Or, jusqu'alors, le Gouvernement a manqué d'ambition suffisamment. Le Président Macron a estimé tour à tour que l'on ne pouvait pas parler de crise migratoire et que l'immigration constituait une chance. Son discours a, par la suite, changé, mais les actes ne sont toujours pas là Vous avez manqué d'ambition sur les expulsions. Vous n'avez pas souhaité revenir sur le délit de séjour illégal. En 2018, vous avez étendu le regroupement familial- réunification familiale aux frères et soeurs de réfugiés mineurs, augmentant l'arrivée d'étrangers par ce biais, comme l'a rappelé notre collègue Henri Leroy. Vous n'avez pas fait grand-chose pour les mariages de complaisance.

Vous avez refusé le contrôle aux frontières, sauf au début de la crise sanitaire où vous avez retrouvé la notion de frontières. Fallait-il en arriver là ? Vous avez refusé de conditionner l'aide publique au développement à la délivrance des laissez-passer consulaires. Vous avez refusé la proposition du Sénat concernant la révocation du statut de réfugié pour les personnes condamnées pour apologie du terrorisme. le renforcement des peines complémentaires d'interdiction du territoire pour les étrangers en situation irrégulière qui commettent certains crimes et délits graves. Vous avez refusé d'aggraver les peines pour les trafiquants d'êtres humains. Vous avez refusé que tout rejet définitif d'une demande d'asile d'une demande d'asile vaille obligation définitive de quitter le territoire français. Vous avez refusé d'inscrire les demandes d'asile dans les pays d'origine, comme l'a rappelé Stéphane Le Rudulier. La réalité est que vous êtes liés à des textes supranationaux qui vous empêchent de lutter contre l'immigration de masse. Je pense à la Convention européenne des droits de l'homme.

Nous pourrions aussi évoquer le pacte de Marrakech. Au moment où la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne, pourquoi ne pas renégocier ou suspendre l'application de certaines directives de l'Union européenne ? Le débat que nous avons eu cet après-midi est, hélas, bien fidèle aux précédents. Le résultat, c'est 2 millions d'étrangers en plus durant votre quinquennat, ce qui fait souffrir les migrants mal accueillis et mal intégrés, mais aussi des Français qui se sentent dépossédés et malheureux de cette situation.

La séance est reprise. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée l'élaborer un texte sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants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

l'initiative du groupe Union Centriste, le Sénat a créé une mission d'information sur les conditions de la vie étudiante. J'avais formulé cette demande au mois de décembre 2019, soit quelques semaines avant la crise de la covid. En effet, comme certains observateurs de la vie étudiante, nous étions préoccupés par la précarisation qui touchait depuis plusieurs mois un nombre grandissant d'étudiants. Pour des questions de calendrier, cette mission d'information s'est déroulée au premier semestre de 2021, alors que la crise sanitaire avait entretemps durement touché notre pays, singulièrement le milieu étudiant. La crise de la covid n'a pas créé le mal-être de certains étudiants. Elle l'a amplifié, elle l'a surtout rendu public. L'opinion a alors découvert que la période des études supérieures était pour certains un chemin semé d'embûches : difficulté de boucler les fins de mois, conditions de logement dégradées et coûteuses, accès aux soins compliqué, alimentation insuffisante, etc. Autant de difficultés qui peuvent affecter les étudiants. Pour certains, la réussite des études devient un défi dès lors que le milieu que le milieu familial n'est pas en mesure d'apporter l'aide nécessaire. Notre modèle républicain d'égalité des chances est pour ceux-là fortement altéré. Les images révélées par la crise sanitaire d'étudiants faisant la queue aux Restos du Coeur pour se nourrir ou isolés dans des chambres d'étudiants trop petites sont le résultat en fait d'un triple manquement. l'augmentation continue du nombre d'étudiants non anticipée depuis plusieurs années principalement à l'université, entre 20 000 et 35 000 étudiants supplémentaires chaque année, s'est faite au détriment d'un accueil qualitatif des étudiants. étudiants. Ensuite, les politiques d'accompagnement à la réussite étudiante n'ont pas été prioritaires et n'ont pas fait l'objet d'efforts budgétaires suffisants pour apporter des solutions satisfaisantes aux situations de détresse. Enfin, la population étudiante est peu connue et ses difficultés sont insuffisamment analysées. Malgré le travail de qualité de l'Observatoire national de la vie étudiante, la connaissance que nous avons d'elles est insuffisante à l'échelon national comme au sein de chaque établissement universitaire. Quel est le nombre d'étudiants dans la précarité : 10 %, 15 %, 20 %, plus ? Personne ne le sait. Pourtant, comment ne pas penser que les difficultés de revenu, de logement, de santé sont l'une des causes majeures de l'échec élevé en première année de licence ? C'est dans ce contexte et avec ces questions que la mission d'information a mené son travail pendant plus de quatre mois sous la présidence de Pierre Ouzoulias, que je tiens à remercier non seulement de sa connaissance du secteur, mais aussi du souci qu'il a eu de favoriser un climat de travail consensuel, qui a permis un vote à l'unanimité du rapport d'information et des propositions qui fondent cette proposition de résolution. Quelles sont ces propositions ? Faute de temps, je ne peux toutes les présenter, mais je m'arrêterai quelques instants sur les principales. Elles s'articulent autour de quatre axes : privilégier l'ancrage territorial de l'enseignement supérieur, tirer les conséquences de la crise pour améliorer la condition étudiante,

nous avons tous constaté l'engagement des collectivités territoriales auprès des étudiants. Nous savons également l'importance de l'ancrage local des établissements d'enseignement supérieur au travers des relations qu'ils entretiennent avec les collectivités territoriales, les entreprises et le milieu associatif. Ces relations concourent, entre autres, à favoriser l'accès des étudiants aux stages et à renforcer l'attractivité de nos territoires. Il nous semble donc nécessaire d'intégrer les problématiques d'enseignement supérieur et de leur localisation dans le cadre des politiques d'aménagement de nos territoires. Développer une offre de proximité est un levier d'amélioration de la qualité de vie des étudiants. Nous préconisons une conception territorialisée et diversifiée des cycles universitaires permettant, par exemple, de réaliser un premier cycle dans un établissement de proximité, de taille restreinte, qui favorise un accompagnement personnalisé et évite l'éloignement familial. En quelque sorte, il s'agit de mettre fin au phénomène de métropolisation qui a poussé depuis des années à investir massivement dans de grands centres universitaires. L'ancrage territorial passe également par une offre de logements étudiants adaptée. On le sait, le logement constitue un problème majeur pour un grand nombre d'étudiants. Aujourd'hui, en France, il manque près de 250 000 logements étudiants. Si de multiples plans pour accélérer la construction ont été mis en place, ils ne l'ont pas toujours été de manière efficace et n'ont pas atteint leur cible.

Nous proposons donc d'intégrer pleinement les collectivités dans les politiques de construction des logements étudiants en territorialisant et contractualisant les objectifs avec elles. la prise en compte des spécificités de nos territoires est nécessaire, tout comme la participation de nos collectivités pour proposer une offre pertinente. Au-delà de l'importance du maillage et des politiques territoriales, la crise sanitaire

sur les actions de services de médecine préventive et de promotion de la santé, dont le champ d'action est très limité et dont les moyens demeurent insuffisants. À titre d'exemple, il y avait au début de la crise un équivalent temps plein, ou ETP, d'infirmière pour 10 000 étudiants, un ETP de médecin pour 16 000 étudiants et un ETP de psychologue pour 30 000 étudiants. Le taux de couverture est donc faible, alors que seulement un étudiant sur quatre déclare consulter un service médical durant son parcours universitaire. La crise sanitaire a mis en lumière l'insuffisance et les limites de ce système et a contribué à l'émergence de nouveaux besoins, notamment en matière d'accompagnement psychologique et de prise en charge des frais de santé. Du point de vue de la prévention psychologique, par exemple, il existe seulement dix-huit bureaux d'aide psychologique universitaire (BAPU) en France et certaines agglomérations comme Bordeaux ou Lyon n'en disposent pas. Nous appelons donc à dynamiser sensiblement l'offre de services de santé universitaires par un renforcement des réseaux avec les médecines de ville ou hospitalière, à renforcer l'accompagnement psychologique des étudiants en prolongeant l'accès gratuit aux soins psychologiques et à résoudre les difficultés d'affiliation qui compromettent la protection sociale de certains étudiants ultramarins. la crise sanitaire a mis en évidence la nécessité de garantir un meilleur accompagnement des étudiants. En la matière, elle a montré le rôle clé des établissements universitaires, notamment en matière alimentaire. Je vous rappelle qu'un quart des étudiants dont les difficultés financières se sont aggravées pendant le premier confinement ont déclaré ne pas toujours avoir pu manger à leur faim pour des raisons financières. En conséquence, nous invitons à prolonger le dispositif du repas à un euro dans les restaurants universitaires pour les étudiants boursiers et à faire en sorte que les étudiants aient accès, dans tous les territoires, des oeuvres universitaires et scolaires, les Crous. Au-delà des aides et du soutien financier, il convient de repenser notre rapport à l'emploi étudiant. Même s'il renvoie à une grande diversité de situations, il concourt nécessairement à l'amélioration de la condition de vie étudiante. L'exercice d'une activité peut néanmoins devenir un problème si elle entre en concurrence avec les études. Il est donc nécessaire d'identifier les étudiants pour lesquels la charge de travail liée à cet emploi est susceptible de nuire à la réussite universitaire et de leur offrir un accompagnement personnalisé.

Ces deux dernières années ont aggravé les difficultés financières des étudiants et une grande partie d'entre eux déclaraient ne pas avoir assez d'argent pour couvrir leurs besoins. Je tiens tout d'abord à saluer le travail et l'implication exceptionnels des associations étudiantes durant la crise sanitaire. Elles méritent d'être soutenues. le soutien financier repose essentiellement sur les aides publiques, qui sont constituées pour l'essentiel des bourses et des aides au logement. J'appelle particulièrement votre attention sur la question des bourses. Il y a en effet beaucoup à dire sur les échelons et les effets de seuils. De plus, les bourses ne prennent pas en compte la notion de pouvoir d'achat et la réalité des dépenses liées à la vie étudiante. En fonction de l'implantation géographique ou encore du coût du logement, l'impact sur le pouvoir d'achat n'est pas le même. Nous recommandons donc d'instaurer le calcul d'un « reste à charge » après la prise en compte des dépenses obligatoires pour mieux cibler les étudiants qui ont besoin d'une aide supplémentaire. Nous ne pouvons que regretter que la réforme des bourses pourtant annoncée par le Président de la République n'ait toujours pas été réalisée. Elle semble avoir été abandonnée, n'étant semble-t-il pas jugée prioritaire par Bercy. Quel message, alors que l'État a pourtant trouvé ces derniers mois l'argent nécessaire pour lutter contre les effets de la crise sanitaire ! Je terminerai en soulignant deux autres propositions complémentaires à la réforme des bourses : d'une part, la mise en place d'un dispositif de guichet unique en matière d'aides sociales, d'autre part, l'élaboration et la généralisation d'outils au sein des établissements universitaires pour cibler et assurer l'accompagnement des étudiants ayant un besoin spécifique. Voilà quelques-unes des propositions que nous avons formulées. Veuillez conclure, cher collègue. Elles sont des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les étudiants.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui, résultat des travaux de la mission d'information sur les conditions de vie étudiante en France, fait un constat clair et incontestable : la pandémie, qui nous touche tous depuis deux ans, a frappé de plein fouet notre jeunesse. Ce constat, nous le partageons entièrement. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera cette proposition de résolution. Au-delà des formules consensuelles de ce texte, qui ont permis de rassembler des signatures émanant de toutes les travées de notre assemblée, il me paraît indispensable de dire qu'il y a aujourd'hui urgence à agir pour remédier aux maux qui touchent les étudiants de France

Face à cette réalité, l'aveuglement et le déni du Gouvernement constituent une violence supplémentaire infligée à la jeunesse de France. Dans leur rapport annuel 2020-2021, les Restos du Coeur nous alertent : la moitié des personnes accueillies ont moins de 25 ans

Nous avons tous été saisis d'effroi devant ces files interminables d'étudiants attendant de recevoir une aide alimentaire partout en France, l'année dernière. Beaucoup de jeunes se retrouvent aujourd'hui encore sans filet de sécurité durant leurs études. de cette jeunesse que nous voyons s'enfoncer dans la précarité, nous ne pouvons rester les bras ballants en déplorant de voir une génération sacrifiée. C'est la raison pour laquelle nous défendons, comme nous l'avions fait en 2021 à l'Assemblée nationale, l'instauration d'un « minimum jeunesse », qui passerait notamment par l'extension du RSA au moins de 25 ans. Ce revenu de base pour les jeunes est une proposition de bon sens, d'ailleurs soutenue par deux tiers des Français, qui permettrait de répondre immédiatement à l'urgence sociale concernant notre jeunesse. Ne nous y trompons pas, si la crise liée à la pandémie a amplifié les difficultés rencontrées par les étudiants, elle n'a fait que mettre en exergue les problèmes structurels auxquels l'université française doit faire face depuis beaucoup trop longtemps. La précarisation des étudiants de France, c'est aussi le résultat de son sous-financement. Les moyens alloués à nos universités ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur incombe ! Le Conseil d'analyse économique pointait récemment que le niveau de dépense publique par étudiant est en baisse depuis plusieurs années. Par ailleurs, tandis que les effectifs étudiants ont augmenté de 20 % à l'université ces dix dernières années, le nombre d'enseignants a quant à lui diminué de 2 %. s'ajoutent de très fortes disparités entre cursus : 11 000 euros par étudiant pour un cycle de licence en lettres et sciences humaines, contre 60 000 euros pour un cursus en école d'ingénieurs ; une moyenne de 9 enseignants-chercheurs pour 100 étudiants en école d'ingénieurs, contre 3,5 en licence de sciences humaines. nos étudiants souffrent plus que dans de nombreux autres pays- je peux en témoigner en tant que parlementaire des Français de l'étranger -, c'est aussi en raison de cette exception française d'un système à deux vitesses, grandes écoles et universités, qui favorise les premières au détriment des secondes. Outre qu'il engendre entre-soi et reproduction sociale, ce système favorise une sous-dotation endémique de l'université. Est ainsi créée une concurrence déloyale au profit des plus nantis, ce qui aboutit à un manque de reconnaissance des formations universitaires, terreau rendu fertile pour nourrir la détresse des étudiants les plus vulnérables. N'oublions jamais que prendre soin de notre jeunesse, c'est prendre soin de l'avenir de notre pays. C'est aussi se donner les moyens d'affronter les défis climatiques, économiques et démocratiques qui sont devant nous.

la crise sanitaire qui frappe notre pays et le monde depuis maintenant deux ans aura bouleversé nos vies à bien des égards. Elle aura aussi été un électrochoc pour les 2,8 millions d'étudiants en France, un révélateur de la précarité dans laquelle un grand nombre d'entre eux se trouvent. Elle aura ainsi mis en lumière un malaise certain auquel il nous faut répondre. Comment ne pas comprendre ce malaise, lorsque l'on voit ces étudiants faire la queue pour recevoir une aide alimentaire ? Comment ne pas comprendre ce malaise, lorsque l'on entend les témoignages d'étudiants déprimés, isolés, alors même que l'on a coutume de dire que les années d'études supérieures sont les plus belles de nos vies,

Celle-ci a avant tout permis d'écouter les principaux concernés, en premier lieu les associations d'étudiants, afin de mieux comprendre cette réalité. Elle a également apporté, grâce aux nombreux échanges et déplacements effectués durant près de quatre mois, des pistes de réflexion intéressantes pour répondre aux difficultés que rencontrent les étudiants dans leur quotidien. d'information issu de nos travaux verse donc au débat un certain nombre de propositions sur des thématiques diverses. Je pense à la crise du logement et aux 250 000 logements étudiants qui manquent pour répondre à la demande. Nous proposons notamment de relancer la dynamique de création de logements étudiants sur l'ensemble du territoire en prenant en compte les perspectives d'évolution de la démographie étudiante et le prix local de l'immobilier. Je pense à l'accès aux soins, à la santé psychologique et à l'alimentation, quand nous savons que près d'un étudiant sur deux déclare sauter des repas pendant une semaine de cours. La santé mentale des étudiants, en particulier durant cette période de crise sanitaire, doit également être au coeur de nos préoccupations. Je pense à l'encadrement de l'enseignement à distance, celui-ci ayant parfois montré ses limites pour un certain nombre d'étudiants qui ne disposaient pas d'outils numériques ni même d'un logement adéquat pour étudier dans les meilleures conditions. L'accès aux stages, qui occupent désormais une place centrale dans de nombreux cursus, reste une source de préoccupation pour les étudiants, en particulier pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un réseau à leur disposition. Il s'agit pourtant d'un enjeu majeur, puisque les stages conditionnent souvent l'obtention du diplôme et favorisent une insertion plus rapide sur le marché du travail. À cet égard, le Gouvernement a apporté des réponses concrètes le plan « 1 jeune, 1 solution », doté de 9 milliards d'euros, qui comprend un volet spécifique destiné aux offres de stages. Je pense, enfin, à l'emploi étudiant, puisque quatre étudiants sur dix travaillent en plus de leurs études pour payer leur loyer, rembourser leur prêt étudiant ou tout simplement vivre dans des conditions dignes. Je veux ici saluer le travail de cette mission d'information et l'esprit de consensus de son président, Pierre Ouzoulias, et de son rapporteur, Laurent Lafon, auteur de cette proposition de résolution. Nos travaux démontrent l'intérêt du Sénat pour ces problématiques majeures et notre volonté commune d'y apporter des solutions. Le Gouvernement et la majorité présidentielle sont pleinement conscients des difficultés que rencontrent les étudiants, en particulier durant la crise sanitaire. C'est pourquoi un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour accompagner les étudiants, notamment d'un point de vue financier et sanitaire. Ainsi, le dispositif des « chèques psy » a permis aux étudiants qui en avaient besoin d'aller consulter un psychologue sans avoir à avancer de frais. La mission d'information a d'ailleurs salué ce dispositif et en propose la prolongation. Les repas à un euro pour tous les étudiants, boursiers ou non, furent l'un des outils de lutte contre la précarité alimentaire, que la crise a amplifiée. Le gel des loyers dans les résidences universitaires et le gel des droits d'inscription du dispositif des prêts étudiants garantis par l'État à hauteur de 20 000 euros permet aux étudiants d'emprunter pour financer leurs études, sans apport personnel. La revalorisation des bourses sur critères sociaux est enfin un outil de justice sociale, puisqu'elle permet à des milliers d'étudiants de poursuivre leur cursus dans les meilleures conditions. En tout état de cause, le groupe RDPI soutiendra cette proposition de résolution, qui pose des principes et des recommandations que ses membres partagent pleinement. Son adoption permettra d'envoyer un message fort à l'ensemble des acteurs du monde étudiant et aux étudiants eux-mêmes.

Notre ambition commune consiste à faire en sorte que la « génération covid » et les générations futures puissent s'épanouir dans leurs études, se former et s'insérer durablement sur le marché de l'emploi. Nous voterons donc avec enthousiasme cette proposition de résolution. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, prendre soin de nos jeunes, c'est préparer notre avenir. C'est une évidence pour tous les parents ce devrait l'être pour tous les pays. Investir dans la jeunesse, c'est miser sur l'avenir en stimulant l'excellence qui nous permettra de tenir notre rang. C'est particulièrement vrai pour les étudiants, qui se forment pour participer à un projet de société. Cette période d'études joue un rôle charnière entre deux moments de la vie ; elle cristallise, pour beaucoup, le passage effectif à l'âge adulte. Or, depuis le début de la pandémie, voilà près de deux ans maintenant, beaucoup de nos jeunes ont l'impression d'être passés à côté de leur vie étudiante, si l'on peut dire, comme si le virus leur avait volé ces années qu'on leur promettait si heureuses et si intenses. Ils éprouvent le sentiment d'avoir joué de malchance. Nous connaissons tous des jeunes qui nous ont fait part de cette immense déception. C'est pourquoi je tiens à saluer l'initiative de cette proposition de résolution. Elle a, à mes yeux, l'immense mérite de poser une question fondamentale pour nos travaux : celle de la qualité de vie des étudiants. Indirectement, comme je l'ai dit d'emblée, c'est de l'avenir de notre pays qu'il est en fait question.

Nombre de nos jeunes considèrent déjà- à juste titre, selon moi -que cette période de leur vie a été gâchée par le virus. Pour une large part, le mal est fait, car on ne récupère pas ces années-là.

nous est ainsi donnée de poser un diagnostic lucide sur ce qui constitue la qualité de vie des étudiants. De façon évidente, la crise nous a rappelé que les études ne se résumaient pas à l'absorption de contenus pédagogiques. Tâchons donc, à l'avenir, de nous souvenir que le contact humain avec les professeurs, la convivialité et les échanges intellectuels avec les camarades, la fréquentation des locaux de son école ou de son université, voire le fait d'habiter sur un campus, de vivre là où se crée et se transmet le savoir, d'y faire du sport, bien mise à mal par la pandémie, sont autant d'éléments déterminants pour la qualité de vie des étudiants. Il y a donc une dimension spatiale, physique, des études, qui les ancre dans un territoire, dans une géographie donnée. J'insiste sur ce point, car cette dimension me paraît essentielle aux travaux du Sénat, chambre des territoires. Eh oui, mes chers collègues, on n'est pas étudiant dans le métavers ! Nous sommes tous ici attachés à la dynamisation de nos territoires. Or nous savons aussi l'effet d'entraînement que les lieux de formation, d'études et de recherche ont sur les bassins d'activité.

c'est miser sur une formation, une industrie, un environnement ; c'est accroître l'innovation et l'encadrement au sein même des entreprises locales ; c'est stimuler, demain, un rayonnement de la souveraineté intellectuelle et économique de notre pays. termes, travailler à améliorer la qualité de vie des étudiants, ce n'est pas du tout offrir un confort superflu : c'est investir pour oeuvrer, de façon concrète et opérationnelle, au redressement, à l'indépendance et au rayonnement de notre pays. Très bien ! C'est pourquoi je soutiens plusieurs des recommandations contenues dans cette proposition de résolution. Je pense notamment au dispositif, déjà évoqué, de

euro, lancé par le Gouvernement, qui répond concrètement aux problèmes des étudiants précaires. Je songe enfin à la facilitation du cumul entre études et jobs étudiants, qui contribue aussi à la formation professionnelle. Le deuxième élément de calendrier qui me paraît important, c'est bien évidemment la proximité des prochaines échéances électorales, qui structure largement notre débat public. Dans ce contexte, toute initiative plaçant la qualité de la vie de nos étudiants au coeur des débats est utile. Bien sûr, chacun promouvra des propositions différentes, suivant sa sensibilité politique, mais je crois que nous pouvons tous ici nous accorder sur l'enjeu vital que représente ce sujet pour notre pays. Le troisième et dernier élément de calendrier découle du deuxième : la prochaine rentrée universitaire se fera au cours d'un nouveau quinquennat. Si nous espérons tous qu'elle ne sera pas placée sous le signe de la crise sanitaire, elle sera en tout cas gonflée de nouveaux espoirs, pour certains, de nouvelles craintes, pour d'autres. Ce sera l'occasion de définir de grandes priorités d'action.

tout au long du premier semestre de l'année 2021, notre mission d'information a procédé à une étude approfondie des conditions de la vie étudiante à partir de témoignages d'experts, de représentants d'associations étudiantes et d'acteurs de l'enseignement supérieur. J'ai été très heureuse d'y participer. L'analyse du parcours des étudiants réalisée par notre mission s'est voulue linéaire, s'attachant à relever les obstacles rencontrés par nos jeunes, de leur entrée dans l'enseignement supérieur jusqu'à la préparation de leur insertion professionnelle.

La première rupture est familiale, puisque l'étudiant quitte un environnement affectif connu et protecteur pour un parcours d'études souvent solitaire dans une ville éloignée de celle où il a vécu. La perte de repères induite par cet éloignement géographique et affectif peut être profondément déstabilisante pour ceux qui ont une capacité moindre à s'adapter au changement. La seconde rupture est liée à la nature de la formation choisie. Si un grand nombre d'étudiants font le choix éclairé de la formation dans laquelle ils s'engagent, combien la choisissent par défaut ou par méconnaissance de leurs idéaux professionnels, avec le risque avéré d'un échec, dont ils auront parfois du mal à se remettre ? Pour traiter ces deux problématiques, la mission d'information plaide pour un ancrage renforcé de l'enseignement supérieur dans les territoires. Le choix du campus est fondamental dans le premier cycle d'enseignement supérieur. Pour l'étudiant, la possibilité d'intégrer une formation dans un campus à taille humaine proche de son domicile familial est l'une des conditions de sa réussite académique. À cet égard, l'institut national universitaire d'Albi, dont les formations se répartissent sur quatre sites- Albi, Rodez, Castres et Figeac -, pourrait être érigé en exemple. De taille réduite, il accueille 4 000 étudiants qui, pour 80 % d'entre eux, ont choisi le critère de la proximité géographique de la résidence familiale comme déterminant leur choix de formation. L'implantation de l'université d'accueil dans un environnement familier facilite la transition vers l'enseignement supérieur, voire la conditionne, comme certains experts nous l'ont indiqué. Les étudiants conservent intacts leurs liens familiaux, amicaux ou associatifs. Ils bénéficient aussi d'un accompagnement beaucoup plus aisé et précis que celui dont ils pourraient bénéficier dans des structures universitaires de plus grande taille. C'est pourquoi notre mission d'information préconise de développer un maillage de petites villes universitaires, privilégiant des complémentarités territoriales, à l'image de ce que proposent en Europe l'Italie ou l'Allemagne. La qualité de vie et la réussite des étudiants tiennent par ailleurs beaucoup à l'ancrage territorial des établissements d'enseignement supérieur et à l'engagement des collectivités locales, comme notre mission d'information a pu le constater. Certaines collectivités s'impliquent d'ailleurs directement dans le développement d'une offre locale de formation supérieure. C'est notamment le cas dans le domaine de la santé, avec des formations destinées à pallier le manque de professionnels maîtrisant telle ou telle compétence précise. D'autres s'engagent pour créer les campus de demain, des campus pensés comme des lieux de vie ouverts sur la ville et intégrés à la cité. Il est loin le temps des campus anonymes, désertés par leurs étudiants une fois les enseignements dispensés. Le campus de demain doit offrir des équipements à usage partagé et être un lieu de vie sociale, culturelle et sportive, parfaitement inséré dans le tissu urbain grâce à un effort accru en matière de transports en commun. Les questions d'aménagement du territoire y sont prégnantes, de même que les préoccupations environnementales, d'accessibilité et de logement, comme c'est le cas pour un campus que je connais particulièrement bien, celui de l'université Paris-Saclay. J'ajoute que le lien avec le tissu et les acteurs socio-économiques doit être fort. Pour certaines universités, ce lien est même fondamental et la recherche d'adéquation entre les formations proposées et l'emploi local, destinée à favoriser l'employabilité des étudiants, est une démarche systématisée. Notre mission d'information a constaté que la capacité des établissements à garantir une certaine adéquation entre les parcours de formation et les offres d'emploi, en travaillant avec les acteurs socio-économiques locaux, constituait un facteur très net de différenciation entre universités. Concernant l'université Paris-Saclay, l'interaction entre la recherche et le tissu économique crée les conditions de l'excellence scientifique et de la vitalité entrepreneuriale. Nos étudiants y trouvent un environnement de travail et une qualité de vie particulièrement propices à leur épanouissement et à leur accomplissement personnel et professionnel. Bien entendu, ce modèle ne peut être dupliqué en tout point du territoire, mais il illustre bien la nécessité d'inscrire l'enseignement supérieur au coeur des politiques d'aménagement du territoire en s'appuyant sur l'échelon local, comme le recommande notre mission d'information. Le choix de la proximité pour l'accès à l'enseignement supérieur et l'ancrage territorial des établissements sont parmi les pistes de réflexion les plus crédibles, là où il s'agit d'améliorer les conditions de la vie étudiante en France. Gageons que les travaux et les propositions du Sénat en la matière seront suivis attentivement. Le groupe Les Républicains votera en faveur de cette proposition de résolution. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les étudiants font partie des victimes indirectes, oubliées de la crise sanitaire. Nous savons que cette crise n'a fait que décupler leurs problèmes, tant du point de vue sanitaire et alimentaire qu'en matière d'accès au logement. Au Sénat, nous avons été plusieurs à interpeller le Gouvernement lors des questions d'actualité et à l'occasion de débats. Les réponses apportées n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Je tiens à remercier Laurent Lafon et Pierre Ouzoulias, ainsi que les membres de la mission d'information sur les conditions de la vie étudiante, de leur investissement sur ce sujet essentiel pour l'avenir de la jeunesse de notre pays. Cette proposition de résolution vient conclure notre travail. Elle présente avec acuité les problèmes auxquels sont confrontés les étudiants de notre pays. La fin du confinement et la reprise économique n'ont pas permis à ceux-ci de sortir des difficultés financières et la demande d'aide alimentaire n'a malheureusement pas baissé. Les distributions de vivres se multiplient dans les universités. Les Restos du Coeur ont dû ouvrir un centre dédié à l'université d'Évry. En Gironde, c'est l'équivalent de 220 000 repas qui ont été servis en 2021.

La difficulté à se loger s'accroît d'année en année. Il n'y a pas suffisamment de logements étudiants et les prix du parc locatif privé sont souvent bien trop élevés. La FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, a relevé une augmentation de plus de 5,5 % du montant des loyers à la rentrée 2021 par rapport à 2020. Là encore, nous pouvons compter sur des associations et sur les syndicats étudiants, qui mettent en place des réseaux d'entraide et trouvent, dans la mesure du possible, des logements d'urgence aux étudiants. Reste que de trop nombreux jeunes sont contraints d'abandonner leurs études ou de choisir des filières par défaut, faute de pouvoir se loger et financer leurs études. Les Crous et les universités jouent également un rôle important pour aider les étudiants en difficulté, par le biais d'aides ponctuelles d'urgence,

Tous les acteurs du secteur le disent, la majorité des étudiants qui demandent actuellement des aides ne sont pas boursiers. Madame la ministre, votre gouvernement avait pourtant promis à plusieurs reprises la refonte du système de bourse. Les étudiantes et les étudiants l'attendent toujours. Vous avez jugé cette réforme « trop complexe ». Ne pensez-vous pas qu'il est « complexe » pour les étudiants de dépendre de l'aide alimentaire qu'il s'agit d'une situation infamante pour un pays comme la France ? Les étudiants ne devraient-ils pas n'avoir à se préoccuper que de la réussite de leurs études ? Il faut ajouter à ce triste constat les difficultés d'accès à la santé et le besoin d'accompagnement psychologique, qui s'est fortement accru lors de la crise sanitaire. du groupe Écologiste -Solidarité et Territoires, soutenons évidemment les préconisations de cette proposition de résolution. Cependant, nos attentes pour les étudiants vont plus loin. Nous souhaitons la réforme du système de bourse la création d'une allocation d'autonomie pour tous les étudiants ; l'augmentation significative du nombre de logements étudiants à loyer modéré et la revalorisation des aides au logement ; le rétablissement du ticket à un euro dans les restaurants universitaires pour tous les étudiants, les investissements nécessaires étant de que ceux-ci puissent gérer correctement l'augmentation du nombre d'usagers. Nous souhaitons aussi le recrutement plus massif d'assistantes sociales et de psychologues au sein des Crous et des universités, ainsi qu'une revalorisation de leurs salaires

qui auront des effets positifs sur la vitalité des territoires et amélioreront la qualité de vie des étudiants. Ces mesures ne sont pas « complexes ». Il s'agit non de dépenses inutiles, mais bien d'investissements nécessaires

Elle est symboliquement cosignée par tous les membres du bureau de la mission d'information, donc par tous les groupes politiques du Sénat. Ainsi démontrons-nous sa continuité avec ce travail collectif et exprimons-nous notre accord avec son bilan et ses préconisations. Je remercie Laurent Lafon et le groupe Union Centriste de nous permettre d'en discuter en l'inscrivant à l'ordre du jour des Nul ne peut plus ignorer la profonde dégradation des conditions de vie des étudiants, tant notre pays a été heurté et meurtri par les images de ces jeunes réduits à trouver leur pitance auprès des banques alimentaires. La crise sanitaire n'a été que le point ultime d'une lente déliquescence de leurs moyens de se nourrir, de se loger, de se soigner et, en définitive, d'étudier. les politiques publiques mises en oeuvre depuis au moins deux décennies avaient oublié l'essentiel, que rappelle justement et très simplement cette proposition de résolution : il n'est pas possible d'apprendre le ventre vide, d'apprendre dans la promiscuité d'un logement trop petit, d'apprendre avec une vue mal corrigée, d'apprendre avec un mal de dents non soigné, d'apprendre avec la peur de perdre son emploi précaire quand il apporte tout le revenu. Les étudiants ne sont pas des cerveaux dans lesquels des connaissances sont déversées et que l'on stimule en donnant l'illusion qu'ils participent à une compétition internationale dont les règles les ignorent. Le classement de Shanghai est moins efficace que les Restos du Coeur pour secourir les étudiants ! Notre proposition de résolution relève une évidence coupablement négligée : l'accompagnement personnalisé des étudiants dans toutes leurs activités matérielles est une condition essentielle de leur réussite académique. Notre mission d'information a eu la surprise de constater, à cet égard, que ce sont souvent les petits établissements, éloignés des grandes métropoles, qui ont réussi à proposer aux étudiants les dispositifs d'accompagnement les plus efficaces. Ce résultat est obtenu par la mobilisation exceptionnelle de toutes leurs équipes au service de la réussite des étudiants. Je prends à mon tour, après Laure Darcos, l'exemple de l'institut national universitaire Champollion d'Albi. Son succès est double. Il offre un cursus universitaire à des jeunes issus de la ruralité qui n'auraient eu ni les moyens financiers ni même la volonté de s'inscrire dans une université de taille supérieure et il parvient à les conduire jusqu'à la fin de la licence par un suivi individuel de grande qualité. Son taux de réussite est ainsi l'un des meilleurs de France. Ce travail profite aux étudiants, mais aussi à leurs territoires. Il est donc regrettable que cette excellence républicaine, qui vise la promotion des individus et des collectivités dans lesquelles ils vivent, ne soit pas mieux aidée valorisée., cet exemple vertueux démontre que l'échec en licence n'est pas une fatalité et qu'il est possible de le résorber par des politiques volontaristes adaptées à chaque situation. Affirmons-le avec force : il y a une solution budgétaire, donc politique, au problème de la réussite estudiantine. L'origine des difficultés profondes dont souffrent les universités est unanimement reconnue : c'est le sous-investissement chronique. Le Conseil d'analyse économique, organisme placé auprès du Premier ministre, et la Cour des comptes viennent très récemment de l'analyser sans contredit. Je ne retiens que deux chiffres, déjà cités, de ces bilans affligeants. La dépense intérieure par étudiant baisse inexorablement depuis plus de dix ans et, durant la même période, les effectifs étudiants ont augmenté de 20 %, quand le nombre d'enseignants diminuait de 2 %. Le Conseil d'analyse économique considère que cette dépression budgétaire a des conséquences économiques néfastes sur le marché du travail, la productivité et l'innovation, mais aussi sur la cohésion sociale, car l'université est incapable de corriger les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur. Il estime qu'il faudrait consacrer entre 5 milliards et 8 milliards d'euros supplémentaires par an pour remettre à flot le système universitaire. C'est beaucoup d'argent, mais finalement bien peu pour donner à notre jeunesse des raisons d'espérer dans son avenir et à notre pays une voie pour surmonter les épreuves à venir par l'investissement dans la connaissance et l'engagement républicain renouvelé en faveur de l'émancipation humaine. Je vous remercie

Il nous donne l'occasion de poser un diagnostic sur la vie étudiante grâce à une réflexion dépassant le simple cadre des problématiques liées au quotidien de l'étudiant et à son accompagnement matériel, ou à son parcours d'études. Si la crise sanitaire que nous vivons a mis en lumière la précarité d'une part croissante de nos étudiants, les difficultés structurelles préexistaient. Ces dernières ne disparaîtront pas avec la fin de la pandémie. La question est donc la suivante : quelles perspectives pouvons-nous offrir à nos jeunes pour améliorer leurs conditions de vie et d'études, particulièrement dans le contexte sanitaire actuel, mais également à plus long terme ? La mission d'information a formulé plus d'une cinquantaine de recommandations pour améliorer la condition étudiante. Devant l'augmentation régulière du nombre d'étudiants au cours de la période récente, et face à un système qui est, à certains égards, à bout de souffle, il est urgent d'agir de manière globale. Comme vous l'avez vous-même déclaré, madame la ministre, avec la pandémie, la vie étudiante est sortie de la périphérie des politiques publiques. La première question déterminante est celle du logement. Elle peut conditionner les choix d'orientation du futur étudiant lorsque l'établissement visé implique de quitter le domicile familial. Les conditions dans lesquelles l'étudiant est logé ont aussi des conséquences sur son parcours et sa réussite dans l'enseignement supérieur. Or le constat est sans appel : l'offre de logements en résidences étudiantes, qui s'élève aujourd'hui à 350 000 places, est structurellement insuffisante par rapport à la population étudiante, estimée à 2,7 millions en 2019. Même si ces résidences n'ont pas vocation à accueillir tous les étudiants, les capacités demeurent vraiment insuffisantes. En 2018, le Gouvernement a annoncé un plan visant à construire 60 000 logements étudiants à l'échéance de 2022, ce que nous avions salué à l'époque. Mais les objectifs de ce plan ne sont pas atteints.

Une réflexion pour territorialiser les objectifs de construction de logements étudiants en fonction du nombre d'étudiants et des perspectives d'évolution de cette population doit être amorcée.

Avec le logement, les dépenses d'alimentation constituent la principale charge des étudiants. En fonction de leurs moyens financiers et des charges fixes auxquelles ils ne peuvent se soustraire, les achats de nourriture, essentiels par définition, deviennent une variable d'ajustement : cela les conduit souvent à s'alimenter de mauvaise qualité, ou bien à ne rien manger du tout ! Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire que nous vivons n'arrangent pas la situation, qui perdure donc. Les associations comme les Restos du Coeur alertent sur le sujet depuis 2019 déjà, les moins de 25 ans représentant parfois 50 % de leurs bénéficiaires. Le 1 décembre dernier, les associations d'aide alimentaire étudiantes tiraient de nouveau la sonnette d'alarme sur l'extrême gravité de la situation en formulant le constat suivant : « Les étudiants ont faim. » Dans les files d'attente des épiceries solidaires, les témoignages ressemblent beaucoup à ceux de l'automne 2020. Malgré des efforts importants, un décalage persiste entre l'offre de restauration universitaire et la demande des étudiants. Les principales raisons de ce décalage sont connues, et sont régulièrement pointées du doigt l'éloignement de certains sites ou filières d'enseignement par rapport à l'implantation des structures de restauration ; les délais d'attente dans certains restaurants universitaires ; les contraintes liées à l'emploi du temps des étudiants ; ou encore la faible amplitude horaire d'une grande partie des restaurants universitaires, peu adaptée aux besoins des étudiants. Un dispositif tel que le ticket restaurant étudiant aurait pu atténuer ces disparités. Là encore, c'est par une logique d'approche territoriale qu'il faut raisonner, en favorisant les partenariats entre les réseaux des oeuvres universitaires et scolaires et les acteurs publics et économiques locaux le but est de permettre à chaque étudiant d'avoir accès à une offre de restauration à tarif social. Il me paraît important d'évoquer les aides publiques auxquelles peuvent être éligibles nos étudiants. Elles interviennent souvent en complément d'autres ressources, et peuvent représenter, pour un boursier, jusqu'à la moitié de ses ressources. être évités s'agissant de ces aides. Le premier tient à leur complexité et à leur manque de lisibilité, ce qui les rend « particulièrement difficiles à appréhender pour un public encore jeune et peu habitué aux démarches administratives

Ainsi, je ne peux que souscrire aux recommandations formulées par la mission d'information, à savoir l'expertise du phénomène de non-recours des étudiants aux droits sociaux, l'amélioration de l'accès des étudiants à l'information au moyen d'un portail unique recensant toutes les aides publiques susceptibles d'être attribuées par les différents acteurs et l'évolution vers un dispositif de « guichet unique » en matière d'aides directes. Enfin, il est urgent de revoir notre système de bourses sur critères sociaux, notamment en simplifiant l'architecture des échelons pour atténuer les effets de seuil. Madame la ministre, mes chers collègues, il est nécessaire d'aller vers un ancrage territorial de l'enseignement supérieur, qui doit être inscrit au coeur des politiques d'aménagement du territoire, en s'appuyant sur l'échelon régional. Les étudiants sont un facteur de dynamisme et de transformation, et une richesse pour nos territoires. Pour conclure, je souhaite remercier mes collègues membres de la mission d'information « Conditions de la vie étudiante en France » pour leur travail de fond, et plus particulièrement son président Pierre Ouzoulias

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'augmentation continue du nombre d'étudiants, associée à une situation sanitaire exceptionnelle, a révélé l'urgence d'une nouvelle réflexion sur la vie étudiante. Cette réflexion a été menée au sein de la mission d'information « Conditions de la vie étudiante en France », présidée par notre collègue Pierre Ouzoulias. Le rapport d'information fait au nom de la mission par Laurent Lafon et la proposition de résolution dont nous discutons aujourd'hui,

des étudiants qui arrivent dans l'enseignement supérieur sont très hétérogènes. Dans le cadre de la délégation à la prospective, nous avions entendu M. Olivier Babeau : il préconise une période de propédeutique- pourquoi pas une année ? -afin de permettre aux étudiants de combler leurs lacunes et de renforcer leur autonomie dans le supérieur. Il s'agirait de concevoir un dispositif qui ne léserait pas les étudiants faisant le choix de cette remise à niveau, comme c'est parfois le cas actuellement. Ainsi, en médecine, des étudiants n'ont pu trouver de places en première année à la suite de cette année blanche,

Il existe un grand nombre de structures payantes, des « officines privées » parfois très coûteuses, aidant les étudiants à préparer les travaux dirigés et les examens en parallèle de leurs cours. Un système de tutorat interpromotion permettrait aux étudiants d'améliorer leurs chances de réussite et à leur famille de réaliser des économies. existe déjà dans certains établissements : il serait bon de le généraliser, ce qui permettrait également de renforcer les liens sociaux entre étudiants, liens qui ont été grandement affectés par la généralisation des cours à distance. Il convient donc de s'interroger sur la gratification des tuteurs sous forme de bourses ou de points de bonification. J'aimerais également insister sur le temps de l'inscription dans l'enseignement supérieur. Trop souvent négligé, il constitue pourtant un moment décisif : il faut le mettre à profit pour communiquer aux étudiants toutes les informations utiles sur les aspects de la vie quotidienne dans leur futur établissement,

nous y proposons de lancer une consultation de l'ensemble des acteurs de la vie étudiante afin de préciser le périmètre d'affectation de la contribution. Il s'agit aussi de décider s'il faut pérenniser, ou non, le financement par la CVEC de dispositifs exceptionnels mis en place pendant la crise, notamment l'octroi d'aides financières. Je voudrais aussi évoquer la question de l'ancrage territorial de l'enseignement supérieur dans les grandes villes universitaires et dans les plus petites collectivités territoriales.

De même, l'accueil de doctorants, par exemple, a des retombées très positives permettant de dynamiser certaines filières territoriales. Je terminerai mon propos en citant les campus connectés, qui constituent une véritable opportunité pour les personnes vivant loin des établissements supérieurs. Ils recréent du lien social par l'enseignement à distance. Ce dispositif fonctionne bien, et l'offre de formation gagnerait à être développée sur l'ensemble du territoire. Alors que certaines universités ont choisi de faire cette rentrée en distanciel, restons attentifs à ce que les étudiants traversent cette période d'incertitude dans les meilleures conditions possible. La

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les études de l'Observatoire de la vie étudiante prouvent que les conditions de vie et d'apprentissage ne cessent de se dégrader. Le Gouvernement ne semble toujours pas mesurer la gravité des faits, alors que 21 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté et que 13 % d'entre eux ont déjà eu des pensées suicidaires. Beaucoup essayent, tant bien que mal, d'allier emploi alimentaire et études. Certains revoient leurs objectifs d'études à la baisse, parfois même abandonnent l'université. J'ai une pensée émue pour cet étudiant de 22 ans qui, dans l'impossibilité de faire face à ses multiples difficultés, avait tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu en novembre 2019. Qu'a donc fait le président Emmanuel Macron pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage de la population estudiantine ? Presque rien. Alors que le candidat promettait en 2017 la construction de 60 000 logements universitaires, seuls 16 300 ont été livrés en 2021. C'est pourtant ce poste de dépense qui pèse le plus dans le budget des étudiants. Il est même parfois insurmontable. Pour pallier cette difficulté, une revalorisation des aides au logement était nécessaire. Emmanuel Macron a précisément fait l'inverse, en baissant de 5 euros les APL. Alors que la crise sanitaire exacerbe les difficultés, les étudiants attendaient un geste politique fort du Gouvernement. La mise en place des repas à 1 euro et des aides financières exceptionnelles, souvent excluantes et inadaptées, ne permet pas de répondre à un problème qui est en réalité structurel. Les universités se transforment en centres d'aide sociale face à l'inefficacité de l'action gouvernementale. Centraliser les dispositifs d'aide afin de les rendre accessibles est un objectif primordial : il faut pour cela octroyer des moyens supplémentaires aux Crous, afin qu'ils L'instauration d'un revenu de base, gage d'autonomie et de réussite scolaire, est également une priorité absolue face à un système de bourses devenu obsolète. Je doute que le gouvernement en place nourrisse réellement cette ambition de réforme. Je voterai toutefois pour ce texte,

cette proposition de résolution fait suite aux travaux que nous avons menés dans le cadre de la mission d'information sénatoriale « Conditions de la vie étudiante en France ». Le président Laurent Lafon et le groupe Union Centriste nous donnent l'occasion d'y revenir aujourd'hui, et je les en remercie. Notre pays compte 3 millions d'étudiants : ce chiffre a plus que doublé depuis les années 1980. Il prouve que la France a relevé le défi de la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Mais cette bonne nouvelle doit être relativisée par le taux d'échec en première année et en premier cycle, les mauvaises orientations, les réorientations, et surtout par la précarité que subissent de nombreux jeunes durant leur cursus. nous amener à nous interroger sur l'insuffisance des moyens mobilisés au service de cette jeunesse, mais également sur la pertinence des schémas dans lesquels la politique d'enseignement supérieur s'inscrit et se déploie.

après l'ère et l'essor des grands pôles d'excellence situés dans les métropoles, de réfléchir à la place et au rôle que pourraient jouer les petites et moyennes villes dans l'accueil de formations supérieures innovantes. Vous le savez, ces villes jouent déjà un rôle dans l'équilibre du territoire : elles constituent une armature territoriale précieuse pour notre pays. Elles offrent également des conditions d'hébergement intéressantes, puisque les loyers y sont plus accessibles que dans les grandes villes françaises. Mais il ne suffit pas de créer un premier cycle d'études dans une petite ou moyenne ville pour considérer que l'État a rempli sa mission. Il faut également des enseignements de qualité, des enseignants de renommée nationale, mais aussi tous les services et les équipements que le réseau des Crous déploie avec une efficacité remarquable. Je pense bien sûr aux restaurants universitaires, et à l'offre sociale, sportive et culturelle. Cette proposition de résolution est un plaidoyer en faveur de la coexistence d'une offre diversifiée comme mes collègues du groupe socialiste, j'ai la conviction que les pôles d'excellence universitaire dans les métropoles, qui répondent aux critères des classements internationaux, peuvent et doivent coexister avec des structures de proximité qui soient également attractives et performantes. Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur le logement étudiant, qui est un vrai défi pour beaucoup de jeunes. Accéder à un logement de qualité à un loyer abordable est une gageure pour de nombreux Français. Pour les étudiants, cela ressemble à un véritable parcours du combattant. J'ai la chance de venir d'un territoire où le Crous- celui de Montpellier -est particulièrement dynamique en matière de rénovation et de construction de logements. Je veux rendre hommage à ses directeurs successifs Philippe Prost et Pierre Richter. Ce résultat est la conséquence d'un travail partenarial engagé depuis quinze ans avec les collectivités locales : la région Occitanie, la métropole de Montpellier, les communes et les bailleurs sociaux.

Fort de cette expérience, je vous propose de tendre vers la territorialisation des objectifs de construction de logements. Cela passe par leur inscription systématique dans les contrats de plan État-région

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si les étudiants sont très majoritairement épargnés par les formes graves de contamination au covid-19, ils n'en demeurent pas moins les victimes collatérales d'une crise sanitaire inédite. Parfois reclus loin de leurs proches lors des confinements successifs, souvent privés des emplois étudiants indispensables à leur subsistance dans le cadre de leurs études, ces derniers ont payé un lourd tribut au coronavirus. Toutefois, si la pandémie a contribué à l'aggravation des symptômes du mal-être étudiant, celui-ci n'a rien de nouveau. Au contraire, la situation sanitaire a permis de mettre en lumière le caractère structurel des difficultés rencontrées par les étudiants et les défaillances profondes des politiques étatiques déployées à leur égard. Certes, des mesures conjoncturelles pour leur venir en aide ont été lancées dans le contexte de la pandémie, à l'image des repas à 1 euro dans les restaurants universitaires, ou encore du « chèque psy », mais ces mesures ponctuelles et très circonscrites, pour louables qu'elles soient, ne sont pas à la hauteur des problématiques auxquelles est confrontée notre jeunesse. C'est la raison pour laquelle je salue cette proposition de résolution, qui vient compléter les réflexions déjà menées par la mission d'information sénatoriale sur les conditions de vie étudiante. Lors de nos travaux, nous avions été attristés de découvrir le nombre d'étudiants concernés par des situations de grande précarité et incapables de subvenir à leurs besoins élémentaires. Face à l'allongement des files d'étudiants aux portes des associations de distribution alimentaire, dont il faut ici saluer le travail indispensable, il apparaît primordial de prolonger de toute urgence le dispositif du repas à 1 euro dans les Crous pour les boursiers afin que chacun de ces jeunes puisse manger à sa faim. Mais répondre à l'urgence ne suffit pas. Pour résorber les inégalités, il faut aller plus loin ! C'est pourquoi je me réjouis de la proposition de créer un nouveau statut d'étudiant salarié dans les établissements universitaires eux-mêmes, afin que les étudiants les plus fragiles ne soient plus contraints de choisir entre leur dignité et leur réussite universitaire. Par ailleurs, la lutte contre les inégalités entre les étudiants doit commencer dès l'entrée à l'université. Je considère qu'une diversification des critères d'entrée est indispensable, comme c'est le cas dans d'autres pays européens.

Au-delà de la question des inégalités, en tant que rapporteure de la mission d'information sur la contribution de vie étudiante et de campus aux côtés de notre collègue Bernard Fialaire, j'ai eu l'occasion de mesurer l'importance de la lisibilité et du traçage de l'utilisation des aides publiques pour les étudiants. Notamment destinée à favoriser l'accueil culturel et sportif des étudiants, la CVEC pourrait, et devrait, contribuer à renforcer le financement des associations étudiantes fragilisées par la crise sanitaire.

Je souhaiterais enfin dire un mot de l'adaptation numérique intervenue dans les universités à la faveur de la crise sanitaire. Si la diversification des outils digitaux permet désormais d'assumer une dématérialisation des enseignements, cette possibilité doit être développée, mais elle doit demeurer une exception. Espaces de vie en commun, d'émulation et de bouillonnement intellectuel, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent demeurer les épicentres de la vie étudiante. Il est donc vital de donner la priorité, chaque fois que cela est possible, au présentiel sur le distanciel, afin d'éviter une dégradation dans l'accompagnement, la formation, mais aussi le bien-être psychologique des étudiants, alors même que les mesures de confinement nous ont permis de mesurer les conséquences psychologiques délétères de l'isolement sur la santé mentale de nombreux jeunes.

Si la pandémie a creusé certaines inégalités en dégradant en premier lieu la situation des jeunes et des travailleurs précaires, elle a aussi aggravé la précarité étudiante et en a fait un enjeu central du débat public. Mais la crise sanitaire que nous continuons à traverser a surtout été un révélateur et un amplificateur de difficultés déjà existantes de la vie étudiante, qu'il s'agisse de la santé, du logement ou de l'alimentation. Si la précarité étudiante n'est pas née avec le confinement, elle s'est en revanche fortement aggravée avec lui. Parmi de nombreux points, je voudrais ici évoquer la problématique spécifique de la santé mentale de nos étudiants. Leur situation a connu une évolution assez singulière. L'état de la pandémie à la rentrée permettait d'envisager des enseignements sur site, mais la hausse du taux de circulation du virus a nécessité la mise en place de nouveaux confinements, avec une fermeture des établissements d'enseignement supérieur et une généralisation de l'enseignement à distance. Quand d'autres secteurs connaissaient un retour relatif à la normale, les conditions d'enseignement uniquement en distanciel et l'isolement qui en résulte ont eu des incidences sur le ressenti et le bien-être de nos étudiants, altérant parfois leur santé mentale. Comme le montre

S'il est vrai qu'une plus grande attention accordée à la santé mentale dans le débat public peut favoriser les déclarations des étudiants sur le sujet et donc rendre visible une détresse jusqu'alors ignorée, il n'en reste pas moins que ces résultats démontrent une dégradation effective de la santé mentale de nos étudiants. Les conditions singulières de cette dernière année, pendant laquelle les étudiants se sont vu imposer davantage de restrictions que le reste de la population, ont accentué cette tendance. Quatre catégories d'étudiants apparaissent particulièrement fragiles : les étudiants en difficulté financière, les étudiants étrangers, les étudiants les plus âgés et les étudiantes. Ces fragilités se traduisent par un recours accru à des structures dédiées ou à des professionnels de santé pour des problèmes émotifs, nerveux, psychologiques ou de comportement au cours des douze mois. On regrettera que le dispositif spécifique du « chèque psy », mis en place en février 2021, ne soit que très peu utilisé par les étudiants.

Confinés loin de leurs familles, les étudiants ultramarins ont été particulièrement touchés par la pandémie. Aux difficultés psychologiques liées à la solitude s'est ajouté, comme pour de nombreux autres étudiants, le découragement lié aux cours en visioconférence et à des équipements informatiques souvent insuffisants, a débouché sur une perte de motivation importante et sur une tentation répandue de décrochage. Mes chers collègues, la santé mentale des étudiants est devenue un enjeu social crucial quand on sait que 75 % des troubles psychiatriques et psychologiques débutent avant l'âge de 24 ans. Les études correspondent à une période de changement dans la vie de l'individu et les étudiants sont souvent soumis à plusieurs formes de pressions, qu'elles concernent la réussite scolaire, les difficultés financières ou l'intégration sociale. Il est donc primordial de tirer les enseignements de la crise sanitaire sur leur santé. Dynamiser l'offre de services de santé universitaires, mais aussi mieux accompagner psychologiquement nos étudiants avec la prolongation de l'accès gratuit, sur prescription médicale, aux aides psychologiques me paraît donc essentiel, pour que leur souffrance psychologique cesse enfin d'être une fatalité. La parole

évidemment dommage que le programme 231 n'ait pas pu être examiné dans cet hémicycle lors de la discussion budgétaire- je sais que je ne suis pas la seule à le penser ici. Je salue le travail nourri réalisé par le président Lafon, le sénateur Ouzoulias et l'ensemble des sénatrices et sénateurs qui ont participé à la mission d'information « Conditions de la vie étudiante en France », un sujet qui est l'un des fils rouges de mon action depuis bientôt cinq ans. ans. Depuis 2017, je n'ai eu de cesse de rappeler que la vie étudiante est un facteur déterminant de la réussite des étudiants. En effet, mon action s'est toujours portée vers une approche globale des étudiants. Aussi, je me réjouis de constater que nous convergeons, puisque l'essentiel des sujets mis en avant dans votre proposition de résolution a d'ores et déjà été pris en compte par le Gouvernement. Comme je l'avais annoncé le 9 juillet dernier, la rentrée 2021 s'est déroulée en présentiel. Cette reprise a été un véritable succès collectif, que nous devons non seulement aux équipes des établissements d'enseignement supérieur et des Crous,

Cette rentrée en présence était particulièrement attendue et demandée, notamment dans le texte de cette proposition de résolution, car jamais le tout numérique en solitaire n'a formé ni ne formera un projet pédagogique.

à son territoire de vie. À cette fin, nous avons consacré 160 millions d'euros pour engager ce travail de modernisation de l'offre de formation et surtout pour apprécier tout le potentiel du numérique dans la construction des formations.

nous avons pu et nous pouvons aujourd'hui maintenir les examens en présentiel. Je veux également souligner l'immense sens des responsabilités dont ont fait preuve autant les étudiants que les chefs d'établissements et les directeurs de Crous. Au cours du premier trimestre de l'année universitaire, nous avons dénombré une soixantaine de clusters pour 2,7 millions d'étudiants et 300 000 agents, ce qui est bien différent des chiffres que nous avons pu connaître. Les événements festifs, culturels et sportifs ont pu être organisés en début d'année, dans le respect des protocoles et avec l'application du passe sanitaire. Au-delà des enjeux strictement sanitaires, la crise a accentué les difficultés sociales que peuvent rencontrer certains étudiants. Pour y faire face, nous avons relevé d'un montant supérieur à l'inflation les bourses sur critères sociaux, et cela trois années de suite, après des années de stagnation. Nous avons mis en place deux aides exceptionnelles, une première de 200 euros et une seconde ouverte à tous les étudiants boursiers à hauteur de 150 euros. Les fonds d'aides des Crous ont été doublés et leur octroi a été simplifié. Par ailleurs les étudiants boursiers et ceux qui, sans être boursiers, bénéficient d'une aide au logement ont pu toucher l'indemnité inflation de 100 euros annoncée par le Premier ministre. Les étudiants boursiers ont d'ailleurs été les premiers, au début du mois de décembre, à voir cette aide versée sur leur compte. Le produit de la CVEC, 150 millions d'euros par an en moyenne, a été fortement mis à contribution dans les universités pour accompagner socialement les étudiants au moyen de distributions de cartes d'achats ou de fournitures informatiques, mais aussi pour créer des centres de santé.

Je songe aux épiceries sociales et solidaires, aux actions menées au sein des résidences universitaires lors des confinements ou encore aux actions en faveur de la santé mentale avec des projets visant à « aller vers », à repérer et à orienter. Enfin, nous pouvons nous réjouir de disposer dans notre pays d'un réseau des oeuvres étudiantes, les Crous, qui maille l'ensemble des territoires en lien avec les établissements et les collectivités territoriales.

Vous le constatez, voici là encore une recommandation de votre résolution que le Gouvernement a d'ores et déjà mise en oeuvre. Par ailleurs, pour permettre au plus grand nombre d'étudiants d'accéder à ces repas, nous poursuivons la montée en charge des conventionnements entre les Crous et les restaurants administratifs sur tout le territoire. Parce que le projet d'émancipation pour la jeunesse que défend ce Gouvernement est un projet global, j'ai voulu que nous prenions aussi des mesures pour lutter contre la précarité menstruelle, contre le mal-être des étudiants. Depuis février dernier, des distributeurs de protections périodiques gratuites ont été mis en place. De même, nous avons instauré la gratuité de la contraception jusqu'à 25 ans. S'agissant du bien être psychologique, nous savons que la crise a renforcé le mal-être de certains, mais le Gouvernement y a répondu massivement. En moins de six semaines, nous avons mis en place la plateforme « Santé Psy » qui fédère près de 1 800 psychologues en France, pour permettre à tous les étudiants de bénéficier d'un parcours de soins pris en charge jusqu'à huit séances. plateforme, 18 000 étudiants ont bénéficié de près de 120 000 séances. Cela vient en complément de l'action menée par les services de santé universitaire, où j'ai voulu que nous doublions le nombre de psychologues. Au-delà des dispositifs d'aide, c'est également en soutenant comme jamais la reprise économique et le développement des emplois étudiants que le Gouvernement a travaillé à soutenir les étudiants. Au coeur de France Relance, le plan Jeunes annoncé en juillet 2020 par le Premier ministre représente plus de 6 milliards d'euros consacrés à la jeunesse. Nous avons créé et pérennisé 20 000 emplois de tuteurs et ainsi financé autant d'emplois étudiants, pour 3,6 millions d'heures tutorées chaque semestre. Nous avons créé 1 400 emplois de référents dans les cités universitaires, au plus près des étudiants.

sans compter l'impact de la reprise économique, associé au plus faible taux de chômage observé chez les jeunes depuis des décennies. Ces réponses à la crise n'ont en réalité fait que renforcer l'engagement constant du Gouvernement en faveur des étudiants depuis 2017 pour associer l'amélioration des conditions d'études et la réussite académique. Le plan Étudiants doté de 1 milliard d'euros que j'ai présenté en octobre 2017 exprimait déjà cette ambition. Nous avons ouvert l'affiliation automatique de tous les étudiants au régime général de la sécurité sociale, ce qui représente pour eux une économie de 217 euros par an. Sous le précédent quinquennat, la sénatrice Procaccia avait très justement formulé le problème, mais rien n'avait été fait. Le plan Étudiants a aussi permis la création du droit à l'année de césure, la création de licences modulaires fondées sur des blocs de compétences pour mieux articuler l'offre d'enseignement aux réalités territoriales de l'emploi, ou encore la création des bachelors universitaires de technologies en trois ans entièrement tournés vers l'insertion professionnelle, et la possibilité pour les collectivités d'être maintenant partie prenante des contrats d'établissement. Intervenue par vagues successives depuis plusieurs dizaines d'années, ne pouvait constituer une fin en soi si elle impliquait de renoncer dans le même temps à massifier la réussite, et donc à réellement démocratiser l'enseignement supérieur de notre pays. C'était tout l'enjeu de Parcoursup et tout l'objet des « oui si », ces parcours de remédiation et d'accompagnement vers la réussite qui ont été mis en place dans les universités. Force est de constater que ce diagnostic était le bon : en quatre ans, et la L2 ont progressé de plus de 4 points, alors que depuis vingt ans l'échec en licence semblait devenu une fatalité. Je n'ai pas peur de dire que nous avons travaillé, depuis 2017, à une véritable politique de territorialisation de l'enseignement supérieur,

dans le cadre de la mission que le Premier ministre vous avait confiée sur ma proposition. Nous avons également créé des ponts vers l'enseignement supérieur dans tous les territoires. Ce sont 89 campus connectés et 60 campus « coeurs de territoires en zone rurale, qui permettent à chacun d'accéder à l'enseignement supérieur dans un cadre tutoré, en lien avec un établissement d'enseignement supérieur, sur le modèle des meilleures pratiques internationales, notamment celles du Canada. Et cela marche : le taux de réussite est de 70 % dans ces lieux. Territorialiser l'enseignement supérieur était aussi au coeur de la réforme des études en santé.

Promouvoir l'enseignement supérieur dans tous les territoires, c'est aussi faire confiance aux modèles en devenir. Il y a quelques semaines, je me suis rendue à Mayotte et à cette occasion, le Gouvernement a annoncé la transformation prochaine du

au-delà des désaccords et des divergences politiques, donne parfois quitus au Gouvernement de son travail et de ce qui a été réalisé. Naturellement, il reste beaucoup à faire afin de répondre à la demande croissante de formation supérieure, et cela tout au long de la vie. Nous avons déjà travaillé à engager la fin du sous-financement de nos universités et de nos établissements d'enseignement supérieur. Comme chacun le sait, plus de 1 milliard d'euros de moyens supplémentaires pérennes ont été consolidés chaque année dans le budget des universités. La programmation de la recherche, France Relance et France 2030 viendront prolonger ce qui avait été engagé dès 2017 dans le plan Étudiants. Le Président de la République, comme l'ensemble du Gouvernement et comme vous- j'en suis sincèrement ravie, croyez-le pense fermement que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dessinent l'avenir de ce pays, à travers sa jeunesse, dans l'ensemble des territoires. Sachez que vous pourrez toujours compter sur moi pour défendre cette vision. La discussion

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis très heureux que notre Haute Assemblée puisse aujourd'hui se pencher sur cette proposition de résolution, rédigée avec mon collègue Jean-Pierre Moga. Notre ambition est d'identifier les freins au développement de l'agrivoltaïsme en France. Une première question se pose : qu'y a-t-il derrière ce terme ? Nous considérons que l'agrivoltaïsme peut participer à relever les nombreux défis qui se présentent à l'agriculture française défense de notre souveraineté alimentaire, le maintien et la reconquête de la biodiversité, mais également la production d'énergies renouvelables. En effet, le secteur agricole assure aujourd'hui près de 20 % de la production française d'énergies renouvelables, et 13 % de la production photovoltaïque nationale. les 437 000 exploitations agricoles françaises, près de 50 000 sont déjà impliquées dans la production d'énergies renouvelables. Le nombre d'exploitations agricoles engagées dans la production d'énergie décarbonée pourrait d'ailleurs tripler d'ici à 2030. Toutefois, il existe un risque : celui des conflits d'usage et du « grignotage » du foncier agricole. Produire de l'énergie sur une parcelle agricole ne doit pas remettre en question la vocation première des terres fertiles, celle de nourrir. Il nous faut prendre ce risque de conflit d'usage au sérieux afin de protéger les terres agricoles de l'artificialisation des sols. Notre proposition de résolution s'inscrit dans cet engagement, alors que notre pays a déjà perdu le quart de sa surface agricole au cours des cinquante dernières années. Nous estimons que l'agrivoltaïsme peut et doit permettre de surmonter un tel risque, en associant les deux productions sans consommer de terres agricoles, dans un objectif de coproduction, de non-artificialisation des sols et d'écologie territoriale concrète. L'agriculture bénéficiera de nombreuses synergies résultant de cette association entre agriculture et énergie, car s'il y a bien une compatibilité entre les deux productions, l'ambition de l'agrivoltaïsme tel que nous le concevons dans ce texte est d'optimiser avant tout la production agricole, afin d'améliorer le rendement des cultures, d'apporter un complément de revenus aux agriculteurs et d'adapter notre agriculture au changement climatique. L'agrivoltaïsme stress hydrique, avec une réduction de l'évapotranspiration l'été et une baisse de 12 % à 37 % de la consommation d'eau ; celle du stress lumineux, avec une meilleure photosynthèse du stress thermique lors d'épisodes de fortes chaleurs, en réduisant les brûlures sur les feuilles, fruits et branches, ou lors d'épisodes de gelées printanières, avec un écart de température moyen de 2 degrés déterminant pour les cultures. En résumé, la production agricole peut être améliorée par cette double production et les synergies constatées. Une seconde question se pose : quelles sont les ambitions de cette proposition de résolution pour la filière agrivoltaïque ? Au cours de nos échanges avec les acteurs de la filière, nous avons identifié trois freins, tant législatifs que réglementaires, qui entravent le bon développement de cette association agricole vertueuse. Premièrement, nous avons constaté l'absence criante de définition de l'agrivoltaïsme. En raison de technologies diverses et de besoins hétérogènes, force est de constater que l'agrivoltaïsme ne dispose d'aucun référentiel commun et souffre d'un manque de définition.

Nous nous sommes ainsi rendu compte que le point de départ de toute réflexion dans le domaine consistait à se mettre d'accord sur la signification de ce terme et sur l'exigence qui devait lui être associée. Nous sommes enfin d'avis qu'une définition claire et rigoureuse permettra de soutenir le déploiement des projets les plus ambitieux, d'accompagner les agriculteurs et d'engendrer un cercle vertueux avec des conséquences en cascade, notamment sur les appels d'offres- j'y reviendrai car il est inacceptable que des projets sans aucune vision agricole se revendiquent de l'agrivoltaïsme. Deuxièmement, nous estimons que l'agrivoltaïsme manque de leviers pour se développer. Parmi les incitations, les principales concernent les tarifs d'achat de l'énergie déterminés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Celle-ci met en oeuvre des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables en instruisant des appels d'offres, actuellement décomposés entre le le photovoltaïque au sol, pour une enveloppe de 10 gigawatts sur la période 2021-2026, le photovoltaïque sur bâtiments, pour une enveloppe de 5,5 gigawatts, et le photovoltaïque innovant, pour une enveloppe de seulement 0,7 gigawatt.

les investissements sont élevés pour les exploitants agricoles, avec une rentabilité économique inégale et incertaine, qui ne se confirme qu'après plusieurs années. Ces coûts microéconomiques sont paralysants et constituent un frein à l'essor des énergies renouvelables dans le secteur agricole. Dès lors, partant de ces constats, les auteurs du présent texte formulent quatre propositions. La première consiste à inscrire une définition de l'agrivoltaïsme au sein du code de l'énergie. Nous la voulons claire, ambitieuse, et reprenant la définition des appels d'offres de la CRE « des installations permettant de coupler sur une même parcelle agricole une production électrique d'origine photovoltaïque secondaire à une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement ».

l'agrivoltaïsme. Les panneaux posés sur les hangars agricoles ne seraient pas concernés par cette nouvelle famille d'appels d'offres. La troisième proposition consiste à rendre éligibles les exploitations agricoles pratiquant l'agrivoltaïsme aux financements européens de la politique agricole commune En effet, un arrêté du 9 octobre 2015 limite les « activités non agricoles » sur les surfaces agricoles, empêchant dès lors l'agrivoltaïsme de bénéficier des aides de la PAC.

Enfin, la quatrième et dernière proposition porte sur les pratiques de compensation agricole collective. Nous estimons que ces pratiques, qu'il s'agisse d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs, d'aides à la prévention et au redressement d'exploitations agricoles en difficulté ou encore d'aides à l'acquisition de matériel agricole, sont vertueuses en ce qu'elles permettent à l'énergie photovoltaïque de soutenir l'agriculture. Elles sont également symptomatiques de l'état d'esprit d'une filière dont le projet est assurément agricole. Or il subsiste de trop grandes divergences entre les territoires

représente un secteur stratégique pour le développement des énergies renouvelables en France. Cette coproduction est vertueuse en raison de nombreuses synergies agroéconomiques, démontrées notamment par les études de l'Inrae

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui est présentée par ses auteurs comme ayant pour objectif de reconnaître l'agrivoltaïsme, « qui devient et se constitue comme une filière en soi, faisant émerger une nouvelle figure au sein du monde agricole : les énergiculteurs en croit cette proposition de résolution, des obstacles persistants freineraient le développement de cette filière. C'est, en effet, une filière en devenir, qui doit encore se structurer, mais c'est aussi une filière qui, malgré sa fraîcheur, se porte bien.

projets sont portés par des collectifs d'agriculteurs et soutenus par des sociétés privées. Ils sont également accompagnés, de manière plus ou moins volontariste, par les communes. Cette filière s'inscrit donc dans nos priorités nationales,

Dans ce contexte, la municipalité de Joux-la-Ville, située à 16 kilomètres au nord d'Avallon, est engagée avec détermination dans le développement des énergies renouvelables. Elle a ainsi décidé d'aller plus loin, en travaillant avec un collectif d'exploitants agricoles et la société Innergex, sur un projet photovoltaïque innovant.

Conformément aux délibérations du conseil municipal de Joux-la-Ville, la création d'un fonds de reconversion agricole est prévue. Ce fonds, abondé par le développeur privé, sera consacré à la mise en place de nouvelles pratiques agricoles. En effet, la municipalité a souhaité qu'un hectare de panneaux installés se traduise par un hectare de « cultures nouvelles ». Des réflexions sont ainsi en cours à propos d'un projet collectif de production, de transformation et de commercialisation de plantes aromatiques et médicinales.

En effet, le chiffre d'affaires par hectare d'une surface d'agrivoltaïsme représente un ordre de grandeur bien supérieur au montant des aides à l'hectare de la PAC.

que les bénéfices de l'agriculteur ne proviennent que de l'énergie photovoltaïque et non plus de sa production agricole. Enfin, il est nécessaire d'éviter tout dévoiement de cette pratique. Sur ce sujet, sans doute sera-t-il nécessaire de développer un modèle d'agrivoltaïsme plus vertueux, grâce à des panneaux intelligents qui s'orientent en fonction de la

lorsque ses modules photovoltaïques sont situés sur une même surface de parcelle qu'une production agricole et qu'ils influencent celle-ci en apportant directement un des services listés ci-après adaptation au changement climatique, accès à une protection contre les aléas climatiques et de prédation ou encore amélioration du bien-être animal et de l'agronomie,

Madame la présidente, monsieur le ministre,

les terres sont de moins en moins nombreuses et l'artificialisation abusive des sols est un défi majeur auquel nous devons répondre d'urgence. il est crucial de poursuivre l'effort de développement des énergies renouvelables, notamment solaires, pour atteindre un mix énergétique permettant notre indépendance et la neutralité carbone. L'agrivoltaïsme s'inscrit dans cette double problématique, à la fois agricole et énergétique. C'est un secteur complexe, parce qu'il se situe à la confluence de ces domaines, dont les priorités ne sont pas toujours identiques.

La production d'énergies renouvelables sur une exploitation agricole va dans le sens de la transition écologique et de l'écologie pragmatique de progrès que défend le groupe Les Indépendants. Elle facilite la production d'une énergie verte, qui peut bénéficier tant à l'exploitant qu'au réseau pour lequel l'énergie sera rachetée. En introduisant la notion d'agrivoltaïsme, cette proposition de résolution met en lumière la possibilité, pour les agriculteurs, de valoriser leur production agricole grâce à la production énergétique. Ces installations permettent à ces derniers de contenir leurs coûts de production, en créant et en revendant de l'énergie, mais également d'optimiser leurs cultures. Ce faisant, elles contribuent aussi aux objectifs nationaux de zéro artificialisation des sols à l'horizon de 2030 et de capacités solaires installées J'ai pu le constater dans mon territoire, des exemples concrets ont déjà vu le jour. La société GreenYellow a signé, en juillet 2020, un accord de coopération avec ArcelorMittal Projects Exosun, pour la réalisation d'une première centrale sur grande culture en Haute-Garonne. Les travaux ont commencé et cette centrale offrira bientôt une production de 2 637 mégawattheures par an, ce qui équivaut à la consommation de 735 foyers. Bien sûr, les retours d'expérience seront cruciaux.

La première priorité est de s'entendre sur une définition légale de cette activité, à inscrire dans le code de l'énergie. Cette étape est essentielle pour pouvoir reconnaître ce secteur et encourager l'émergence d'une filière en France.

La crise sanitaire nous a rappelé la nécessité de maintenir notre souveraineté alimentaire. La France doit rester indépendante et capable de produire ce qu'elle consomme. l'agriculture doit être l'activité principale et la production d'énergie l'activité secondaire. L'objectif est l'optimisation de la production agricole et non la production énergétique. Ce n'est que dans ce cadre clair que les dérives seront évitées. De la définition de l'agrivoltaïsme découlent les questions de financement et d'investissement spécifique. La Commission de régulation de l'énergie aura un rôle à jouer des appels d'offres particuliers, qui restent pour l'instant marginaux. L'agrivoltaïsme n'étant pas compatible avec tous les territoires, toutes les cultures ou tous les élevages, il sera fondamental que ces appels d'offres prennent en compte les impacts fonciers potentiels et encouragent les technologies les plus vertueuses. La possibilité d'un financement par le biais de la PAC doit aussi être explorée. Enfin, comme avec toutes les activités de production d'énergies renouvelables, nous allons nous trouver confrontés au problème du stockage. Certaines solutions existantes paraissent parfaitement adaptées aux projets d'agrivoltaïsme. Je pense notamment au, qui permet de produire de l'hydrogène et de le stocker.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord saluer l'initiative de cette proposition de résolution, qui vise à allier l'agriculture et la transition énergétique, prise par Jean-François Longeot, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et plusieurs de ses collègues. Ce débat permet de rappeler l'importance de l'agriculture pour la production alimentaire ainsi que son rôle dans la transition énergétique, pour décarboner notre économie. Aujourd'hui, l'agriculture contribue à hauteur d'un cinquième à la production d'énergies renouvelables en France, lesquelles représentent 20 % du mix énergétique. Le secteur agricole, grâce à la biomasse, à la méthanisation, au photovoltaïque et à l'éolien, dispose des atouts nécessaires pour apporter une contribution capitale. À titre d'exemple, en Mayenne- terre d'élevage par excellence -, le potentiel de méthanisation permettrait d'assurer l'autonomie énergétique du département. Pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, la France doit accélérer le déploiement des installations solaires et mener de front la transition énergétique et la défense de sa souveraineté alimentaire. L'agrivoltaïsme consiste en l'installation de panneaux solaires sur- et non à la place Cette pratique permet de protéger les cultures tout en produisant de l'énergie renouvelable. Le développement de l'agrivoltaïsme est une solution pour préserver les surfaces agricoles tout en atteignant les objectifs de la transition énergétique. C'est indispensable, car nos agriculteurs, déjà touchés régulièrement par des prix de vente trop faibles et les effets du dérèglement climatique, doivent aussi affronter un défi propre à ce siècle, celui de la pénurie des terres agricoles. J'ajoute qu'il faut être très attentif à ce que la diversification des revenus des agriculteurs n'empiète pas sur la production alimentaire. Cette proposition de résolution « esquisse des solutions pour lever ces freins afin de donner un soutien aux projets d'agrivoltaïsme qui pourraient faire de notre pays un modèle en la matière Les freins identifiés sont au nombre de trois : le manque de définition, le manque de leviers et le manque de financement. Comme l'écrivent les auteurs de la proposition de résolution dans leur exposé des motifs, les « projets agrivoltaïques ne sont pas éligibles aux aides de la politique agricole commune [ ...] en raison de l'aspect innovant de cette double culture. Or, eu égard à ses nombreux avantages agricoles, à la création de valeur dans les territoires ruraux ainsi [qu'à] sa participation [à] la production d'énergie renouvelable, elle est pleinement légitime à en bénéficier ». La PAC doit donc évoluer. Profitons, monsieur le ministre, de la présidence française de l'Union européenne pour mettre ce thème en débat. Nous avons, en Europe, une agriculture qui supporte les normes les plus exigeantes, donc tout ce que nous ferons contre notre agriculture, nous le ferons aussi contre l'écologie, qui est une des priorités du XXI siècle. Il me semble également indispensable de mettre en place des

J'ajoute que le monde agricole a besoin de plus de formation, de conseil et d'accompagnement, afin de mieux préparer les agriculteurs à opérer cette transition agroécologique. Il faut aussi encourager les complémentarités entre l'agriculture et le solaire photovoltaïque. La crise sanitaire a montré que l'agriculture française était résiliente et qu'elle assumait ses responsabilités. Elle peut produire une alimentation saine pour tous et pour tous les budgets. Faisons-lui confiance et maintenons la diversité de nos agricultures sur le territoire national. Il faut accompagner l'ensemble des agricultures pour

et toutes les possibilités de déploiement doivent être étudiées. En ce sens, l'agrivoltaïsme peut jouer un rôle pivot dans cette production énergétique, en conjuguant production agricole et production électrique, tout en préservant, bien sûr, le principe fort de non-artificialisation des sols et de maintien des surfaces agricoles.

Si nous manquons encore de recul et de retours d'expérience sur cette filière, il est clair que celle-ci semble disposer, de prime abord, d'un certain nombre d'atouts : outre la ressource d'énergie verte, nous pouvons citer le soutien économique apporté aux exploitations et la protection contre les aléas liés au dérèglement climatique. C'est pourquoi nous rejoignons les auteurs de cette proposition de résolution sur les principales recommandations formulées pour favoriser son déploiement. Toutefois, pour nous, écologistes, plusieurs principes doivent primer. Tout d'abord, nous soutenons un agrivoltaïsme contrôlé et dont les pratiques sont encadrées. Nous souhaitons la mise en place d'un cadre juridique clair, pour que les projets réellement vertueux et efficaces voient le jour, afin de nous prémunir ainsi des effets indésirables d'un développement non maîtrisé, à l'instar du déploiement de certaines unités de méthanisation. types d'installations agrivoltaïques ont déjà démontré leur inefficacité, comme les panneaux solaires installés sur les toits de serres maraîchères, qui ne permettent pas une vraie production agricole. Autre principe majeur : les cultures alimentaires doivent bien évidemment toujours prévaloir par rapport à la production d'énergie, un des principaux enjeux de l'agriculture pour les années à venir étant notre souveraineté alimentaire. point essentiel : les installations photovoltaïques doivent d'abord s'implanter sur des espaces déjà artificialisés ou, en complément avec l'agrivoltaïsme, sur des terres peu fertiles, en déprise agricole, qui pourraient être remobilisées. Les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) réalisent, tous les cinq ans, un inventaire des friches agricoles, un travail important et utile pour identifier les terres où l'agrivoltaïsme peut être vertueux. Enfin, nous entendons qu'il existe un risque de spéculation foncière quant à la transmission des fermes. En effet, l'agrivoltaïsme peut inciter des agriculteurs retraités à ne pas vendre leurs exploitations pour conserver cette activité. C'est pourquoi la rémunération de l'agriculteur ne doit pas devenir une rente découplée de l'activité agricole. Oui, l'agrivoltaïsme peut être une possibilité de développement dans les territoires agricoles en déprise, mais des garde-fous sont nécessaires pour limiter l'envolée des prix du foncier, pour interdire l'installation sur des terres productives, pour ne pas remettre en cause la pérennité du métier d'agriculteur. De plus, les installations ne doivent pas entraîner une diminution de la production agricole, elles doivent au contraire la conforter. La question de l'implantation des panneaux- écartement et hauteur -est à cet égard essentielle. Quant aux préconisations formulées dans cette proposition de résolution, permettez-moi d'y revenir quelques instants. La nécessité de définir l'agrivoltaïsme est tout à fait justifiée : les enjeux de biodiversité et de non-artificialisation des terres doivent être des objectifs centraux.

La question de la compatibilité avec le droit européen se pose. Sur ce point, nous sommes preneurs des éléments que vous pourrez nous apporter, monsieur le ministre. Je conclus en rappelant que les retours d'expérience sur ces projets sont assez faibles. Il nous paraît donc judicieux de prendre davantage de recul afin d'avoir une base plus solide de bonnes pratiques et de données exploitables et de légiférer en conséquence, à l'issue d'une période exploratoire. Ces enjeux soulignent également un peu plus la nécessité d'une planification, par un service public, des énergies renouvelables, afin d'éviter des déploiements anarchiques, guidés uniquement par le profit et donc mal acceptés par nos concitoyens.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens, dans un premier temps, à remercier les auteurs de cette proposition de résolution sur le développement de l'agrivoltaïsme. En effet, ce sujet soulève de multiples questions, dont nous avons eu l'occasion de débattre au cours des derniers mois revenu des agriculteurs, préservation du foncier agricole, développement des énergies renouvelables et évolution de notre mix énergétique, un des outils permettant d'atténuer les effets du changement climatique. En ce sens, ce sujet n'est pas anodin, car il soulève de nombreuses interrogations liées à la question de la multifonctionnalité de l'agriculture et de la vocation des agriculteurs à fournir à la société des biens autres qu'alimentaires. En effet, agriculture et énergie sont fortement liées. D'une part, l'agriculture est un secteur clef dans la transition énergétique et climatique. Si elle est fortement émettrice de gaz à effet de serre, environ 20 % de la production d'énergies renouvelables française en est issue. À cet égard, À cet égard, l'énergie en agriculture ne peut plus être considérée comme un enjeu secondaire. D'autre part, les agriculteurs sont les premiers touchés par le changement climatique, par la perte de biodiversité et par l'appauvrissement des sols.

de la grêle -ou encore de permettre de réduire la consommation d'eau. Toutefois, si le secteur agricole a toute sa place dans la production d'énergie, il n'en demeure pas moins qu'il faut veiller à ne pas engendrer des conflits d'usage de la terre et une concurrence entre production alimentaire et production non alimentaire. Cela peut être le cas pour le photovoltaïque sur les terres agricoles, présenté à la fois comme une énergie renouvelable rentable, comme un complément de revenu pour les agriculteurs et comme une activité compatible avec l'activité agricole, et qui a connu une progression rapide au cours des dernières années, mais qui suscite de nombreuses résistances. En effet, alors que 18 % des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté et qu'un tiers seulement de leurs revenus est issu de l'agriculture, l'énergie solaire a des airs de nouvel « or vert » pour les agriculteurs, qui ont de plus en plus de mal à vivre de leur activité. Or le risque est grand de voir se développer des fermes photovoltaïques qui stériliseraient les surfaces agricoles et entraîneraient un renchérissement du foncier agricole, de nombreux exploitants accueillant sur leurs terrains des dispositifs photovoltaïques en contrepartie d'un loyer d'un loyer généreux. Pour autant, toutes les formes de production solaire ne sont pas à exclure. Ainsi, pour l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'agrivoltaïsme est une façon d'éviter les conflits d'usage et il s'intègre dans le système agricole et alimentaire dans son ensemble. C'est pourquoi il est indispensable, comme le soulignent les auteurs de cette proposition de résolution, de donner une définition précise de l'agrivoltaïsme, afin de le distinguer du photovoltaïque au sol. De même, il est indispensable de rappeler que la production alimentaire doit rester la priorité et que le développement du photovoltaïque doit se faire au service de la production agricole. C'est le cas du photovoltaïque innovant. C'est pourquoi il convient de mieux cibler les aides en faveur de ce mode de production énergétique plus respectueux de la priorité agricole, tout en encadrant strictement les surfaces de production solaire et les loyers proposés aux agriculteurs, afin que la part du revenu tiré de la production énergétique ne soit pas disproportionnée par rapport à celle du revenu tiré de la production agricole. La question du revenu paysan ne se résoudra pas par la multiplication des revenus complémentaires, voire de substitution. Comme vous le savez, monsieur le ministre, ce débat continuera de nous animer.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, défense de notre souveraineté alimentaire, réforme de l'assurance récolte, préservation de la biodiversité ou encore non-artificialisation des sols : l'agriculture se trouve assurément au coeur de la transition écologique. Elle est à la croisée des enjeux climatiques et énergétiques. Elle jouera un rôle de plus en plus important dans la production d'énergies renouvelables, comme l'a pertinemment souligné l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans à la production d'énergie dans l'agriculture. D'ici à 2050, la production d'énergies renouvelables du secteur agricole sera multipliée par trois. Toutefois, l'essor des énergies renouvelables dans l'agriculture ne doit pas se faire au détriment de la production alimentaire. Toute ambiguïté doit être levée : il s'agit, avec ce texte, de mettre la production d'énergie au service de la production agricole, et non de faire

et développé dans notre pays. En effet, en conciliant cette double production agricole et photovoltaïque sur une même parcelle et en visant des synergies permettant d'améliorer la production agricole, l'agrivoltaïsme constitue une ressource incontournable pour la réussite des immenses et nombreuses transitions qui s'imposent à notre monde agricole. Ne nous trompons pas, l'objectif premier de l'agrivoltaïsme est agricole. L'association des deux productions apporte plusieurs services à l'agriculture des services écologiques, tout d'abord, en préservant la biodiversité ; des services agroéconomiques, ensuite, en réduisant à la fois le stress hydrique, avec une diminution de la consommation d'eau de 12 % à 37 % en fonction des cultures, et et le stress thermique, en favorisant une meilleure photosynthèse, et en permettant une protection accrue contre les épisodes météorologiques.

Certains viticulteurs ou pruniculteurs du Lot-et-Garonne ont même tout perdu. Si l'agrivoltaïsme ne peut contrer ces épisodes de gelées printanières, il peut en atténuer les effets. il est très complémentaire de la réforme de l'assurance récolte que nous examinerons prochainement.

L'agrivoltaïsme permet ainsi d'optimiser la production agricole, d'améliorer sa compétitivité, de la rendre plus résiliente. Il permet surtout de garantir la vocation agricole des sols concernés.

Ce n'est ni le positionnement ni la philosophie des auteurs de la présente proposition de résolution, qui cherchent, au contraire, à enclencher une dynamique vertueuse permettant de concilier deux productions essentielles, d'apporter un complément de revenus aux agriculteurs et,, de créer de la valeur économique, énergétique et écologique dans les territoires ruraux. Nos échanges avec les acteurs de la filière nous ont permis d'identifier trois principaux freins au développement de l'agrivoltaïsme et de formuler quatre propositions.

manque de leviers permettant d'accélérer la dynamique de déploiement de l'agrivoltaïsme en France les appels d'offres de la CRE ; enfin, manque de financements et incompatibilité des structures agrivoltaïques avec les financements européens de la PAC.

Depuis 2014, les projets de travaux d'ouvrages et d'aménagements susceptibles d'avoir des incidences sur la consommation de foncier agricole font l'objet d'une étude préalable définissant des mesures de compensation collective agricole. Ces mesures sont de plusieurs natures : d'une part, elles visent à reconstituer du potentiel agricole la réhabilitation des friches ou la remise à disposition de parcelles non agricoles d'autre part, elles tendent à mettre en place un projet local de développement agricole au moyen d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs ou à l'acquisition de matériel agricole. Dès lors, monsieur le ministre, le Gouvernement souhaite-t-il s'emparer de cette proposition de résolution pour favoriser le développement de l'agrivoltaïsme en France ? Qu'en est-il des annonces attendues sur cette question depuis plusieurs mois ? Le groupe Union Centriste soutiendra bien évidemment cette proposition de résolution. Il se félicite

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) fixe un objectif de 35,1 à 44 gigawatts de capacité photovoltaïque installée en 2028. Le respect de cette trajectoire suppose de tripler, voire de quadrupler, la superficie consacrée à l'implantation de ces projets. Bien que la production énergétique ne soit pas la première cause de l'artificialisation des sols dans notre pays, l'essor de ce secteur ne doit pas se faire au détriment des sols naturels et de la production alimentaire, laquelle doit rester prioritaire en zone agricole, comme le souligne d'emblée la première phrase de l'exposé des motifs de la présente proposition de résolution. Les contestations qui émergent autour des projets d'installation d'énergies renouvelables ne frappent pas uniquement les éoliennes ou les méthaniseurs. Les conflits d'usage s'amplifient sur le terrain en ce qui concerne le photovoltaïque, en particulier les centrales au sol, qui accaparent les terres agricoles, ce qui soulève des inquiétudes légitimes.

raison d'une synergie de fonctionnement entre les deux systèmes. La production agricole serait même optimisée grâce à l'installation d'ombrières pilotables avec un recours possible à l'intelligence artificielle. Outre sa faible emprise au sol, l'agrivoltaïsme permettrait d'apporter un complément de revenu aux agriculteurs. Sur le papier, cette solution apparaît très intéressante. Dans les faits, on ne peut faire l'impasse sur les risques de détournement des terres de leur vocation agricole et d'accaparement par des exploitations toujours plus importantes. Cela ne doit pas être minimisé : dans certains territoires, on a assisté au développement de serres dotées de panneaux avec une activité agricole réduite ou inexistante. Il est donc indispensable de renforcer le contrôle et de ces projets afin de vérifier qu'ils correspondent bien à la définition de l'agrivoltaïsme que les pouvoirs publics voudraient promouvoir. La création d'un label « agroénergie », comme le préconisait, en 2020, le rapport de notre ancien collègue Roland Courteau et du député Jean-Luc Fugit, au nom de l'Opecst, pourrait constituer une piste afin de faire le tri entre les projets.

Les loyers versés par les énergéticiens dépassent souvent trois à quatre fois les prix des fermages. Oui à la diversification des revenus des agriculteurs ; non à leur remplacement par des rémunérations provenant d'activités annexes. Aussi Aussi faudrait-il instaurer un seuil correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires. Il faut certes une définition, comme le proposent les auteurs de la proposition de résolution, mais aussi un encadrement. Or la proposition de résolution demande au Gouvernement de « lever les freins législatifs et réglementaires », sans préciser les points de blocage qu'elle voudrait voir disparaître. Si je ne suis pas opposé à l'agrivoltaïsme en soi, je ne

Aussi, il est préférable de favoriser le photovoltaïsme sur les toits des bâtiments, quels qu'ils soient, plutôt qu'au sol. Ne faisons pas reposer la responsabilité de la production énergétique sur les terres agricoles dont 88 hectares disparaissent chaque jour en France. Mobilisons davantage les gisements photovoltaïques potentiels sur les friches ou les zones déjà artificialisées.

dans nos exploitations agricoles et les enjeux qui y sont associés. L'actualité de ces derniers mois, particulièrement marquée par les questions énergétiques, nous incite plus que jamais à accélérer la transition énergétique.

Ce défi de premier plan ne doit pas nous faire perdre de vue un autre enjeu majeur, celui de la préservation de la vocation nourricière des terres agricoles. L'exposé des motifs de cette proposition de loi rappelle à juste titre, dès sa première ligne, que « l'agriculture a pour mission principale la production alimentaire

». Aussi, en tant que législateurs, nous devons veiller à protéger à tout prix l'agriculture nourricière de cette compétition, qui ne peut que tourner à son désavantage et dont on constate déjà les premiers effets délétères. Face à l'insuffisance des revenus issus de l'agriculture, de plus en plus d'exploitants se tournent vers la production d'énergie, plus rémunératrice. La tentation est grande, quand on sait que le loyer versé pour une installation solaire peut être dix fois plus élevé que ce que rapporte la terre à un exploitant. Cette mise en concurrence participe, en outre, d'une spéculation sur le prix du foncier agricole et accentue les difficultés d'installation, dans un contexte de doublement du prix des terres agricoles en vingt ans et de raréfaction des terres disponibles. Face à ces constats que je

La jurisprudence, qui repose sur un arrêt du Conseil d'État de 2019, autorise ainsi les projets photovoltaïques sur des terres agricoles tant qu'il existe une production agricole, qu'elle soit principale ou accessoire. L'état actuel du droit est donc peu protecteur pour notre agriculture. À ce stade, mes chers collègues, si la définition retenue dans l'exposé des motifs était volontairement tronquée ou s'il s'agissait d'une omission. Selon la définition en vigueur à la CRE, la synergie de fonctionnement entre production agricole et production électrique doit être « démontrable

résolution, vous citez les bénéfices de l'agrivoltaïsme pour la production agricole, comme la protection face aux épisodes météorologiques, la réduction du stress hydrique, la résilience face au changement climatique ... Ce sont des effets très positifs, mais qui n'existent que pour certains types d'installations, particulièrement innovantes, notamment pour la vigne et les vergers. Or, à l'heure actuelle, comme le rappelle l'excellent article de du 5 décembre dernier, les projets d'agrivoltaïsme « les plus répandus » correspondent à l'installation de panneaux dans des pâturages. On est loin des persiennes pilotées par intelligence artificielle qui permettent d'installer des filets anti-grêle. Aussi, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est tout à fait disposé à soutenir le développement de l'agrivoltaïsme, dès lors qu'il s'agit bien de techniques ayant d'abord pour but d'améliorer la production agricole et non de l'utiliser comme un alibi au profit d'une production plus rentable. S'il était possible d'amender une proposition de résolution, nous vous aurions proposé de reprendre un certain nombre de recommandations permettant d'introduire des garde-fous afin de prévenir toute dérive irréversible sur notre modèle agricole. Pour que ces pratiques innovantes et porteuses d'espoir puissent réellement prospérer, nous devons tout d'abord nous assurer qu'elles ne soient pas « étouffées » par des pratiques moins vertueuses. Aussi, nous aurions pu vous proposer de mettre en place un moratoire sur les projets de centrales photovoltaïques sur des terres agricoles ou naturelles. Autre sujet d'inquiétude, qui tempère les bonnes intentions du texte, les auteurs terminent leur exposé des motifs en résumant l'enjeu de ce texte à l'émergence d'une nouvelle profession agricole : les « énergiculteurs Nous croyons, au contraire, qu'il est plus que jamais nécessaire de défendre les agriculteurs, de leur permettre de vivre de leur travail et non de baisser les bras en actant que seule cette hybridation des métiers peut représenter l'avenir du monde agricole. C'est pourquoi, tout en saluant la démarche de nos collègues qui permet d'ouvrir ce débat, nous nous abstiendrons sur cette proposition de résolution. La parole

Or, comme cela a très justement été rappelé dans un récent rapport du Centre commun de recherche de la Commission européenne, l'empreinte au sol des énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, est très supérieure à celle de l'énergie nucléaire

et les activités économiques, telles que l'agriculture et la sylviculture, mais aussi les bénéfices environnementaux, comme la capacité à produire et la qualité des sols. La mission sénatoriale d'information sur la méthanisation, confiée à nos collègues Daniel Salmon et Pierre Cuypers, a préconisé de soumettre les projets de méthanisation à l'avis préalable des maires. Dans la loi Climat et résilience de 2021, la commission des affaires économiques a prévu l'association préalable des communes littorales aux projets de parcs éoliens en mer et l'information des maires de toute réorganisation des concessions hydroélectriques. C'est donc avec un grand intérêt que j'accueille cette proposition de résolution, dont je remercie chaleureusement les auteurs. Elle vise à promouvoir l'agrivoltaïsme en lui offrant un cadre juridique et en l'intégrant aux appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie et aux fonds de la politique agricole commune. Je souscris pleinement à l'objectif de cette proposition de résolution. L'agrivoltaïsme est bénéfique à nos agriculteurs, qui doivent disposer de toutes les facilités administratives et financières nécessaires. Au-delà de ce texte, je souhaite exposer ma vision de l'agrivoltaïsme. premier lieu, il me paraît essentiel que les activités énergétiques exercées par nos agriculteurs soient accessoires et non principales, facultatives et non obligatoires. En clair, il ne faudrait pas que nos agriculteurs se tournent vers l'énergie, faute de rentabilité suffisante en agriculture. En deuxième lieu, il me semble important que les installations énergétiques respectent des normes rigoureuses sur le plan de l'urbanisme, du patrimoine ou des paysages. Nous sommes très soucieux de l'essor du photovoltaïque, que nous avons promu en zone littorale dans la loi Énergie-climat de 2019, et en zones non artificialisées dans la loi Climat et résilience de 2021. Pour autant, cet essor doit être maîtrisé, territorialisé, qualitatif, respectueux des pouvoirs des maires et des plans des collectivités.

Donner un cadre à l'agrivoltaïsme est utile. À cet égard, je salue les initiatives de droit souple conduites en ce sens : la CRE l'a intégré à ses délibérations ; certains acteurs économiques ont promu de bonnes pratiques en la matière, à l'instar de la charte adoptée par Chambres d'agriculture-France, agricoles (FNSEA) et EDF. Intégrer l'agrivoltaïsme aux appels d'offres ou aux fonds est aussi utile. Pour réussir, cette intégration doit naturellement respecter une neutralité non seulement entre les différentes technologies de production d'énergie solaire, mais aussi entre les procédés de valorisation énergétique

pour lutter contre le dumping environnemental et relocaliser les chaînes de valeur des énergies renouvelables, en France et en Europe. Oui, monsieur le ministre, je pense que nous avons une carte à jouer en agriculture avec les toitures, les serres, les ombrières et toutes les installations de protection du maraîchage, de l'arboriculture ou les bâtiments d'élevage. Nous sommes tous très attachés à ce bilan carbone, puisque nous l'avons

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est difficile de s'opposer à une nécessité qui aura force de loi dans les années à venir : l'agriculture devra participer à la transition énergétique de la France et, pour ce faire, nos exploitations agricoles devront contribuer à la production d'énergies renouvelables. Les auteurs de cette proposition de résolution, que je remercie, nous permettent d'examiner aujourd'hui le développement de l'agrivoltaïsme, lequel pourrait permettre une synthèse entre production agricole et production d'énergie photovoltaïque en fournissant notamment une source de revenus complémentaires aux agriculteurs. C'est également la position des chambres d'agriculture et de commerce. Néanmoins, le développement de l'agrivoltaïsme doit s'accompagner de garanties afin d'éviter tout risque d'anarchie et d'accaparement du foncier, déjà soumis à une pression constante depuis vingt ans, au nom d'un potentiel gain financier.

Autre risque lié au développement de l'agrivoltaïsme : une plus grande artificialisation des sols, alors même que la lutte contre cette dérive est une priorité environnementale pour notre pays. Ce risque est naturellement lié à celui du détournement de l'usage des terres agricoles au profit exclusif du développement des énergies renouvelables.

Cette possibilité peut avoir de graves conséquences sur l'aménagement du territoire. Elle constitue également un problème majeur pour les territoires ruraux, qui se retrouveront dotés d'espaces artificialisés sans activité et sans main-d'oeuvre, l'installation photovoltaïque, une fois réalisée, ne nécessitant que très peu d'investissement humain. Le caractère irréversible de ces installations, finalement plutôt industrielles, sur des terrains « déconstruits », qui ne pourront retourner à leur vocation d'origine, doit également nous alerter et susciter de grandes précautions. Notre pays doit encourager le développement des énergies renouvelables. C'est une priorité indubitable. Toutefois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. À l'instar du foncier agricole, l'agrivoltaïsme doit donc être encadré et contrôlé.

On peut douter néanmoins de son efficacité, une charte n'ayant aucun caractère contraignant. Pour sa part, la Confédération paysanne appelle, dans certains territoires, à un moratoire sur le développement de l'agrivoltaïsme, ce qui rejoint notre position : plein de potentialités, le sujet est également porteur de risques majeurs, qui nécessitent de trouver une position d'équilibre. Combiner développement durable et maintien d'une agriculture vivace est possible, encore faut-il en débattre de manière transparente et réfléchie. Encore une fois, notre agriculture de fermes ne doit pas devenir une agriculture de firmes ni céder aux sirènes d'un capitalisme « court-termiste » aux conséquences désastreuses pour notre souveraineté alimentaire et notre avenir. Diversifier les revenus des agriculteurs est un objectif louable. Si les projets agrivoltaïques en font des « énergiculteurs », on s'engage très clairement sur une pente dangereuse. À cet égard, si les sénateurs socialistes ne s'opposent pas au développement de l'agrivoltaïsme, ils oeuvreront à sa mise en place

tensions. L'agrivoltaïsme, qui désigne des installations permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale tout en favorisant une synergie entre les deux productions, répond à des enjeux d'avenir pour l'agriculture et les agriculteurs. Un rapport du Sénat soulignait déjà, en 2020, que l'agrivoltaïsme constituait une voie « très prometteuse en conciliant production agricole et production d'énergie renouvelable ». En 2022, cette conclusion est toujours valable ; elle est même renforcée par les transformations récentes du secteur agricole. En ce sens, l'agrivoltaïsme est un défi pour le présent et l'avenir du secteur agricole. Il faut l'encourager par des politiques publiques claires. Cette clarté doit être celle de la loi, mais aussi celle de sa mise en oeuvre. La résolution atteint son objectif en posant les fondements nécessaires à une reconnaissance effective

en 2020, la ministre de la transition écologique a voulu limiter les bénéfices de certaines installations en révisant les contrats photovoltaïques conclus en application des arrêtés tarifaires de 2006 et 2010. Certains acteurs de ces contrats En 2021, la même ministre a considérablement facilité l'obtention d'un tarif d'achat, en multipliant par cinq la taille des projets photovoltaïques sur bâtiments ne nécessitant pas d'appel d'offres.

C'est pourquoi les besoins de recalibrage des postes sources et d'adaptation des réseaux doivent faire l'objet d'une attention particulière pour une politique d'aménagement globale. dit -, il est vital que l'agrivoltaïsme ne soit pas dévoyé. La production d'énergie ne doit pas être privilégiée au détriment des besoins agricoles. Le risque est réel, au regard de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui prévoit de doubler les capacités de production d'énergie solaire d'ici à la

En un mot, la production d'énergie doit être au service de l'agriculture et non l'inverse. L'électricité n'est pas une production agricole comme une autre. Pour conclure,

acceptable. Nous devons concilier la production d'énergies renouvelables avec la production alimentaire et la souveraineté agroalimentaire de notre pays, laquelle impose de préserver notre patrimoine foncier affecté à l'agriculture et les activités agricoles.

Cet encadrement est absolument essentiel. D'ailleurs, à la demande du Président de la République, le Gouvernement travaille depuis plusieurs mois à l'élaboration d'une doctrine nationale

donnent lieu à des interprétations très différentes selon les territoires et à une jurisprudence qui peut se révéler extrêmement fluctuante, notamment quant au caractère significatif

donc l'objet de votre proposition de résolution : fixer un cadre national harmonisé allant au-delà des définitions retenues dans le cadre des appels d'offres, afin d'orienter les projets de centrales au sol dans le sens de l'agrivoltaïsme. À cette fin,

trois réunions de concertation avec les organisations professionnelles, en septembre, novembre et décembre, afin de leur présenter diverses orientations et de recueillir leurs avis et préoccupations. Ce faisant, nous cherchons à définir un cadre réglementaire vertueux. Au terme de cette concertation approfondie, il est par exemple